La séance est ouverte, le compte rendu analytique de la précédente conférence a été distribué, je n'ai pas reçu l'observation. Je n'en vois point. Il est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Ministre. Mes chers collègues. Mesdames et messieurs. Cette avec stupeur et tristesse que nous avons appris au coeur de l'été. La disparition si soudaine. Que rien ne pouvait laisser présager de notre collègue Nicole Bricq. Nicole Bricq, les quittés alors que toujours déterminé et infatigable et siéger parmi nous quelques jours plus tôt. Jusqu'au terme de la session extraordinaire. C'est une femme de caractère caractère au sens le plus élevé du terme. Dont la compétence était unanimement reconnu sur tous les bancs de notre assemblée. Elle a voué sa vie entière à son engagement politique en faveur des valeurs auxquelles elle croyait exerçant des responsabilités publiques de Woody vous au sein de son parti, le Parti socialiste. à la fois comme élu local. Comme parlementaire. Né à La Rochefoucauld. Cette fille d'agriculteurs quitta sa Charente natale pour faire des études de droit à Bordeaux où elle obtint une maîtrise de droit privé. Alors qu'elle n'avait que 21 ans est ressorti la nécessité d'un engagement politique. en 1972. Elle adhère au Parti socialiste pour défendre les idées qui lui tiennent à coeur. Lucia Lucia vestiaire par la infidèle. Nicole a toujours aimé la politique. C'était une vocation. Sa détermination sans faille était à ses yeux, le fruit d'une éducation familiale ou 3 valeurs. était au 1er rang. 1er rang. La responsabilité. Au sein du Parti socialiste. Nicole Bricq gravit successivement tous les échelons. Elle fut première secrétaire fédéral, membre du comité directeur, membre du conseil national, secrétaire national chargé de la consommation, délégué national chargé de la fiscalité locale et membre des équipes de campagne au moment des élections présidentielles de Lionel Jospin. L'engagement militant L'engagement militant de Nicole Bricq. Déboucha logiquement en 1986 sur un 1er mandat électif. le conseiller régional d'Île-de-France. Mandat qui devait être suivie de beaucoup d'autres. Son engagement politique, la conduisit aussi à devenir, c'était en 1988 considère technique chargé des relations avec le Parlement et les élus au cabinet de notre ancien collègue Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense et puis elle fut conseillère technique pour les relations avec le Parlement, donc éliminé de Ségolène Royal s'était au ministère de l'environnement en 1992. C'est forte de cette première expérience du monde parlementaire que Nicole Bricq fit son entrée à l'Assemblée nationale, c'était en 1997 comme député de Seine-et-Marne. gens-là, d'abord à la commission de la production et des échanges à la commission des finances, oui, je suis un membre notamment de la mission d'évaluation et de contrôle sur la dépense publique, à se forger à se forger. Une solide compétence en matière de finances publiques et puis l'auteur, c'était en 1988 d'un rapport d'information sur la fiscalité environnementale, suggérant une réforme de la fiscalité au service de l'environnement et un renforcement de l'application du principe pollueur payeur.

c'était en 2004, réélu en 2011 elle siégea sans interruption dans notre assemblée jusqu'à sa nomination au gouvernement, c'est une Dans le cadre de son mandat de sénateur il s'affirma comme une spécialiste incontournable des questions budgétaires et l'une des personnalités les plus éminentes de notre commission des finances le refus, la vice-présidente de 2008 à dominance. J'ai la conviction. Que c'est au Sénat lorsqu'elle devint rapporteur général du Budget, un poste que nous savons tous essentiels que sa vie politique par avoir connu une forme de tournant. à ce moment précis que ses collègues, quelle que soit leur groupe prirent conscience de. Sa rigueur et de ses compétences qui lui permirent d'occuper Les autres fonctions ministérielles. Dans un rapport préalable au débat sur les prélèvements obligatoires, elle restera, si c'était à l'Automne 2011 bilan critique de la politique menée dans ce domaine depuis 2007 a sorti de piste et de propositions pour le quinquennat qui allait venir, notamment sur les niches fiscales et leur suppression et une réforme des modalités de calcul des principaux impôts destiné à qu'accroître leur rendement tout en favorisant les donner une plus grande justice fiscale. C'est au mois de mai 16 très exactement en 2012, à l'issue des élections présidentielles. Que Nicole Bricq fut appelé à exercer des responsabilités gouvernementales. D'abord, ministre de l'écologie, du développement durable, énergie, c'était le 1er gouvernement Jean-Marc Ayrault elle pris les positions conforme à ses convictions en faveur de la protection de l'environnement, souhaitant l'introduction d'une plus grande transparence dans l'attribution des gisements miniers et annonçant la suspension des permis de forage exploratoire d'hydrocarbures au large de la Guyane. Nicole Bricq, qui ensuite, c'était de juin 2012, en mars 2014, ministre du commerce extérieur dans le second gouvernement Jean-Marc Ayrault, fonction qu'elle exerça avec la force de conviction qui va caractériser. Printemps 2014 Nicole Moric revint au Sénat. les gens à nouveau à la commission des finances, et puis à la commission des affaires sociales, Elsa pleinement dans l'exercice de son mandat parlementaire, en particulier à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques présenté par le ministre d'alors, qui portait le nom d'Emmanuel Macron, comme toujours en femme libre et déterminé dans ses engagements, elle fut parmi les premiers parlementaires à soutenir, Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle de 2016, 2017 et parmi les premiers sénateurs a rejoint, Monsieur le Président, le nouveau groupe de la République en marche au sein de notre assemblée.

Elle décrivait alors dans ce qui allait être nous l'ignorions son ultime intervention parmi nous le rôle essentiel du parlementaire, participant à une commission mixte paritaire. Dans les termes que je voudrais rappeler et que nous pourrions je crois tous reprendre à notre compte et je. S'il est un moment privilégié dans la vie d'un parlementaire, c'est bien quand il participe à une commission mixte paritaire, en effet, on dispose pour une fois une entière liberté, on a mis en face de sa responsabilité. Nous savons je poursuis ses mots, nous savons qu'il n'y a pas de mandat impératif pour un parlementaire, il faut choisir l'avoir la meilleure pour arriver. Un compromis positif, tout est dit, me semble-t-il. Sur le bicamérisme. Tout à l'heure, ce riche parcours politique. Nicole Bricq s'était imposé dans chacune de ces fonctions successives, par son travail acharné et ses compétences. à l'occasion d'un entretien donné à La République de Seine-et-Marne, c'était en 2006, elle témoignait en ces termes et handicap qu'elle avait dû à ses yeux, surmonter. C'était une provinciale sans réseau. Sans métier décoller de pouvoir je ne venait pas d'un milieu élevé. Elle ajouté. Je la cite, pour une femme, la politique est un dur combat violent même et qui peut faire peur, il faut avoir une cuirasse, je n'avais pas eu la politique sa vision encore l'opiniâtreté, je n'aurais pas réussi. Oui, forte personnalité, au caractère bien trempé. Elle se faisait observer que je la cite encore d'un homme, on dit qu'il a du caractère. Une femme qu'elle a mauvais caractère. J'ai le mien. Et ici une famille. Passionnément engagé en politique au service de la chose publique et de l'État. Alors chers collègues. Au nom du Sénat tout entier. Je souhaite rendre aujourd'hui dans le très mystique, par delà les mots. Par-delà la tradition rendre un hommage à une parlementaire de 1er plan. Pour l'Intelligence, la compétence, la force de conviction de caractère même été unanimement respecté et faisait honneur à notre assemblée. à ses anciens collègues de la commission des finances. De la commission des affaires sociales assez vous, amis et camarades du groupe socialiste et républicain. Ses amis du groupe, la République en marche, j'exprime au nom du Sénat tout entier notre sympathie Jean-Paul Planchou, son fils Renault à toutes. Sa famille, à ses proches, qui sont ici rassemblés à un certain nombre d'anciens collègues qui ont tenu à être là que je vois ici dans notre tribune demeure, je tiens à leur dire en ce moment de recueillement, là aussi, au-delà des mots. L'émotion du Sénat chacun des du Sénat Nicole Bricq est vraiment présente à cet instant dans notre hémicycle au-delà de nos mémoires. Monsieur le Ministre. Monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, cher Jean-Paul Chartrand non. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous parler cet après-midi et, à travers moi, l'ensemble du gouvernement d'une grande dame qui nous a quitté subitement un samedi d'août Nicole Bricq. J'ai eu la chance de bien connaître Nicole Bricq pour avoir travaillé avec elle lorsqu'elle était ministre du commerce extérieur. Puis quand elle fit le choix de rejoindre le mouvement en marche avec un certain nombre d'entre vous, ici présent. Cette grande dame, que je respecte étant. Avait une voix et un visage singulier. Son visage était le symbole même de la franchise que vous lui connaissiez il exprimait toujours ce qu'elle pensait rien qu'en la regardant, il était assez facile de savoir si le dossier qu'elle avait à traiter lui convenait si la journée était difficile aussi, elle était parvenue à lever les obstacles son humeur n'était jamais voilées n'était jamais, enfin elle était Direct elle aller droit au but, elle pouvait raccrocher au téléphone avant même de dire en revoir et parce que l'essentiel avait été dit son franc- parler, rompez avec les habitudes avec les pratiques convenu, c'était le cas ici, bien sûr, dans cette assemblée qu'elle respectait tant, mais elle ne réservait pas cette franchise au Sénat, elle avait l'habitude de tirs tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, aussi bien dans les enceintes officielles, les comités plus restreints, les réunions avec les militants, ou avec ses collaborateurs, il lui arrivait d'être dur parfois très dur, mais cette exigence elle seule imposer aussi à elle-même. De quoi pendant tout son parcours n'a cessé de nous parler de cette grande dame qui était Nicole Bricq de quoi nous parle-t-elle encore. L'audace. L'audace, c'est le 1er mot qui me vient à l'esprit quand il s'agit de parler de Nicole Bricq l'audace d'une carrière politique qui la voie dès les années 80 devenir première secrétaire de la fédération de Paris au sein du Parti socialiste, l'audace pour une femme de gauche de faire campagne sur une terre de droite et de se faire élire député en 1997 dans la 6ème circonscription de L'audace de porter le projet européen, alors même que l'idée européenne devenait plutôt souvent synonyme de discordes et de défiance et non des noms et de confiance. Ce projet européen était profondément ancrée en elle et elle nous le rappelait souvent l'audace, encore de devenir la première femme, rapporteur général du budget aussi Nicole Bricq était une énorme travail, aucun sujet ne la rebute et même les plus techniques, si cela paraissait compliquée, difficile, ardue, elle se disait : j'y vais. Il a dit aller avec une énergie, une générosité qui a entraîné tout le monde derrière elle. Sa compétence économique était considérable, alors même qu'elle était autodidacte. Elle ne se ménageait pas, jamais elle n'a pas compté les kilomètres, lorsqu'elle était ministre du commerce extérieur. L'audace enfin de rejoindre le mouvement marche dès sa création à l'époque nous n'étions que quelques uns à avoir ce désir fou : lutter contre le sentiment que rien n'était possible que tout avait été tenté, et qu'il était presque déjà trop tard. C'est aussi ce moment de notre histoire collective que nous raconte le parcours de Nicole Bricq, dans les années 80 90, le Parti socialiste, où elle occupe ses premières responsabilités s'adapte aux réalités de l'économie de marché, c'est une social-démocratie qui ne dit pas son nom, qui renvoie, par certains aspects à d'autres évolutions du socialisme en Europe. Nicole Bricq débute au Cérès de Jean-Pierre Chevènement à la gauche du Parti socialiste, elle se rapproche plus tard de Dominique Strauss-Kahn à travers Socialisme et démocratie, dans le but de renforcer le courant réformiste du PS cette volonté réformiste l'amène à rejoindre l'aventure en marche parce qu'elle voyait que ce mouvement proposer un juste équilibre entre la liberté et la protection. La protection sans liberté et stérile la liberté sans protection est intenable. Nous en sommes arrivés à ce constat après des parcours bien différent, mais un point commun : nous rassembler au 1er jour comme nous rassemble encore aujourd'hui une volonté mais qui ne sache jamais lâché, qui est toujours là et que nous sommes, cherchons à mettre en oeuvre désormais aux responsabilités, faire bouger les choses en France et porté le projet européen. Cette passion pour le monde qui vient Nicole Bricq on était l'incarnation oui elle était avec passion, une femme d'avenir. Très tôt, elle a été convaincu de la réalité du réchauffement climatique, de son impact du combat qu'il faut engager pour préserver nos enfants, notre environnement, et celui de nos enfants. Ce en quoi il croyait elle y croyez parce qu'elle avait discuter, échanger, réfléchir. à une époque où se manifestent, si souvent le goût pour le raccourci pour la caricature, elle nous rappelle que l'écoute et puis la délibération est un art si précieux qui font nos modes de vie et nos choix collectifs. Cette force-là, elle a également manifesté lors de son passage au ministère de l'environnement en 2012, elle voulait protéger au large de la Guyane, la faune marine et l'environnement, elle a été jusqu'à dénoncer le code minier. Ce beau souci de l'avenir n'est pas sans une grande liberté. Liberté d'esprit et de liberté d'engagement. Vous le voyez, il y avait à la fois chez Nicole Bricq, son engagement et la façon dont elle s'engager des convictions et un Style. Ce visage et cette voix doivent continuer à nous inspirer. L'un des plus grands héritage que nous laisse cette grande dame et que le futur de la France et dans l'Europe et dans le monde. Que ne seront pas nous même si nous sommes enfermés ou encore inquiets. Que nous serons infidèles, notre histoire, si nous perdons de vue le désir de changer les choses. Vous le savez, Nicole Bricq, était également une femme cultivée éprise de musique classique et de poésie. Au moment de conclure.

Un moment à la fois de mémoire de recueillement et de partage autour de ce que nous avons connues pour certains, nous n'avons pas connu ici avec et autour de Nicole.

Nicole. Conformément à l'usage, je vais suspende la séance pour quelques instants,

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 19 janvier 2017 relatives à la profession de physicien médical et l'ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adoption des dispositions législatives relatives à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, la procédure accélérée a été engagée sur ces 3 textes adoptés par l'Assemblée nationale. Dans la discussion générale commune, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du 1er ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des affaires sociales Madame la rapporteur mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs je viens présenter aujourd'hui devant votre assemblée, au nom de madame la ministre des solidarités et de la Santé, Agnès ans que je représente ici ici 3 projets de loi de ratification d'ordonnances rédigées en application de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Contrairement à une majorité d'entre vous, je n'ai pas été directement impliqué dans les débats parlementaires qui ont conduit à habiliter le précédent gouvernement agir par voie d'ordonnance dans les délais limités et dans les domaines qui vont soumis aujourd'hui mais il paraît néanmoins important de remettre dans leur contexte, chacune des ordonnances qui font l'objet d'un projet de loi de ratification afin d'éclairer nos débats, je m'efforcerai d'être aussi clair que possible dans la présentation de chacun de ces textes dans la description des objectifs qui leur sont associées des conditions dans lesquelles ils ont été élaborés, ainsi que dans leur contenu et dans leurs enjeux propres. Je commencerai en 1er lieu par l'ordonnance relative à la profession de physicien médical, elle reconnaît la profession de physicien médical comme profession de santé, ce qui répond à un des objectifs du plan cancer 2014, 2019, et cela concerne en France une population de 600 radiophysiciens en définissant les conditions d'exercice de la profession de ce soutien médical, ce projet de loi de ratification l'ordonnance parachève un important travail de concertation menée en juin 2016 cette concertation a eu avec les représentants des physiciens médicaux des spécialités médicales concernées telles que l'imagerie médicale, la médecine nucléaire, la radiothérapie et bien entendu avec l'Autorité de sûreté nucléaire. La reconnaissance du métier de physicien médical entendent professions de santé, contribuera à renforcer la qualité et à sécuriser les pratiques dans le domaine de l'utilisation des rayonnements ionisants, il est donc essentiel de donner une définition précise du rôle du physicien médical et de ses missions, l'article 1 de l'ordonnance insère dans le livre de la 4ème partie du code de santé publique, la profession de physicien médical dans le même chapitre que celle de pharmaciens ces 2 professions et entre comment le contrôle de la prescription médicale, contrôle de la dose de rayonnement ionisants pour les premiers et contrôle de la posologie des médicaments pour les seconds. Le livre 2 est désormais intitulé Profession de la pharmacie et de la physique médicale concernant le cadre de la profession de dessin médical ce dernier défini par son expertise au sein d'une équipe pluri-professionnelles qui concerne toute question relative à la physique des rayonnements ou des autres agents physiques dans les applications liées à la thérapie est liée à l'imagerie médicale par les grandes lignes de sa fonction, notamment, la mise au point de la qualité d'image, l'optimisation, l'Exposition au rayonnement et aux autres agents physiques, mais aussi par sa mission essentielle, celle de veiller à ce que les doses radioactives administré au patient soit appropriés à l'état de santé de ce dernier et appropriée au traitement prescrit la déclinaison plus précise des missions et des conditions d'intervention du physicien médical sont renvoyées à un décret au Conseil d'État qui sera prochainement rédigé et concertée. Les articles suivants traite selon un plan commun qui concerne toutes les professions de santé, des conditions d'exercice de la profession de physicien médical des conditions d'enregistrement des diplômes ou encore de l'exercice illégal de la profession, ces différentes dispositions étaient destinées à organiser et à sécuriser l'exercice de la profession et à améliorer la prise en charge des patients, la ministre des solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, je représente ici est à titre personnel, pour des raisons que vous connaissez qui sont liées à son parcours professionnel, particulièrement sensible à ce texte, ce texte permet de comprendre l'intérêt de la profession de physicien médical et de son apport incontestable dans l'amélioration de la qualité des soins, j'en viens à la seconde ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé cette ordonnance dont la ratification est également prévue par le même projet de loi transposant droit interne 3 dispositifs nouveaux, mis en place par une directive européenne de 2013, il s'agit de la carte professionnelle européenne la CPE de l'accès partiel du mécanisme d'alerte, elle introduit par ailleurs au niveau législatif, la procédure pour sécuriser et harmoniser la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens pour les 5 médecins de l'appareillage et pour l'usage du tour de psychothérapeute enfin l'ordonnance supprime ce pour répondre à la demande de la Commission européenne, la condition d'exercice de 3 années imposées aux ressortissants lui lunion européenne pour l'accès en France à une formation de 3ème cycle des études médicales ou pharmaceutique. Je sais, de même que ma collègue et je peux même vous dire qu'elle comprend les inquiétudes que la présentation de ce texte a pu susciter auprès des professionnels de santé au travers de l'introduction des dispositions relatives notamment à l'accès partiel nous avons peut-être revenir en 1er lieu sur les raisons qui ont conduit le gouvernement a présenté ce texte sous cette forme et vous indiquer dans quelles conditions la mise en oeuvre de ce dispositif devra s'opérer la directive communautaire relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du vent, novembre 2013 aurait dû être transposée dans le droit français depuis et au plus tard le 18 janvier 2016. Depuis cette date, la France est exposée à 2 villes motivé de la Commission européenne pour défaut de transposition ce manquement à ses obligations, constitue la dernière étape avant une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne aussi, vous comprendrez mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs que la marge de manoeuvre du gouvernement est de ce fait extrêmement réduite concernant par ailleurs la possibilité qui aurait été ouverte d'exempter l'ensemble des professions de santé, ou certaines d'entre elles du Champ d'application l'accès partiel ce n'était pas juridiquement envisageables : un amendement adopté par votre commission des affaires sociales à procéder à cette exclusion position que le gouvernement ne peut soutenir en effet les dates des différentes analyses juridiques conduite dont celle du Conseil d'État ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une option envisageable au regard du droit et de la jurisprudence communautaire, sauf à prendre un risque politique et juridique important d'exposer la France à une procédure pour défaut de transposition. Je sais que le fait que les autorités françaises n'est pas recouru à cette option a suscité beaucoup d'incompréhension chez de nombreux acteurs, nourrissant l'idée qu'il y aurait eu dans ce cas particulier, une sur transposition de la directive, mais telle n'est pas le cas, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour le rappeler, pour autant, je voudrais vous affirmez au nom de ma collègue Agnès Buzyn qu'elle sera particulièrement vigilante aux conditions de déploiement de l'accès partiel au sein de notre système de santé cette vigilance pourra justifier d'en appeler à la raison impérieuse d'intérêt général, dès lors que l'autorisation d'un professionnel accès partiel fera courir un risque à la qualité et à la sécurité des prises en charge ce risque, il ne peut en effet pas être évacués dans un système où les compétences respectives des professionnels de santé sont complémentaires et articulées entre elles est parfaitement connu des professionnels eux-mêmes et elles-mêmes même comme des usagers du système de santé. La conception comme la mise en oeuvre du processus par lequel chaque dossier déposé par un professionnel en vue d'obtenir une autorisation d'exercice partiel seront dans ce cadre extrêmement rigoureuse en 1er lieu parce que la directive prévoit 3 conditions générales qui doivent nécessairement être remplies, hein, le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son état d'origine, l'activité pour laquelle il sollicite un accès partiel 2 les différences entre l'activité professionnelle exercée et la profession qui pourraient correspondre en France sont aussi importantes que l'application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre demandeurs un cycle complet d'enseignement, et 3 l'activité sollicité en accès partiel peut objectivement être séparé d'autres activités relevant de la profession dite correspondante en France si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, hé bien l'autorisation d'exercice partiel ne pourra pas être délivrée. En 2ème lieu parce que le processus d'examen des dossiers des demandeurs, fait par ailleurs appel à l'expression d'un avis par chaque commission compétente, ainsi que par l'Ordre compétents pour les professions ordre ce second avis non prévues par la directive a été rajoutée par le gouvernement afin de renforcer davantage le processus d'analyse de ces dossiers. En 3ème lieu enfin parce qu'un décret en Conseil d'État va venir préciser les conditions et modalités de mise en oeuvre de la procédure d'instruction, la ministre avait indiqué devant l'Assemblée nationale qu'elle serait extrêmement vigilante à ce que sa rédaction puisse éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers devront être examinées au cas par cas. Ce qui est le cas dans ce projet de texte et qui est actuellement examiné par le Conseil d'État, tout en respectant le droit à la libre circulation des ressortissants européens, le décret dispose en effet que les avis des commissions d'autorisation d'exercice et les ordres seront appelés à émettre porteront notamment dans le but de garantir la qualité et la sécurité des soins d'identification précise et strictement délimité du Champ d'exercice ou des actes que les professionnels sont autorisés à réaliser sous le régime de l'accès partiel la description de l'intégration effective de ces actes dans le processus de soins et leur insu dans ses vents Duel sur la continuité de la prise en charge la lisibilité des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé, comme pour les usagers et les usagères du système de santé toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion de professionnels auquel l'autorisation d'exercice partiel seraient accordé. La rédaction de ce décret et voudrait confie animé par la motivation de garantir la qualité et la sécurité des soins et l'information des professionnels de santé et des usagères et des usagers du système de santé. Par ailleurs, comme ma collègue s'était engagé devant l'Assemblée nationale, elle sollicite la Commission européenne afin d'obtenir une cartographie des professions de santé existantes dans l'Union européenne, la nouveauté induite par le déploiement du mécanisme d'accès à l'exercice au sein des pays de l'Union, justifie en effet que l'on puisse disposer d'un untel, état des lieux permettant d'identifier pour chaque système national de santé, les périmètres d'exercice des professionnels susceptibles de solliciter une reconnaissance d'accès partiel. Et ma collègue, la ministre des solidarités, la santé, m'a demandé de vous rappeler enfin qu'elle sera très attentive au suivi et à l'évaluation qui seront réalisés dans la mise en oeuvre effective de ces dispositifs. Concernant l'ordonnance relative à l'adaptation des dispositions relatives au fonctionnement des ordres de professions de santé, cette 3ème ordonnance a pour objectif de renforcer l'indépendance et l'impartialité des juridiction ordinale ainsi que de faire évoluer les compétences des organes désordre et de l'application par leurs conseils nationaux de la législation relative aux marchés publics, elle intègre un certain nombre de recommandations issues du Conseil d'État, mission d'inspection de juridiction administrative de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des affaires sociales qui ont successivement depuis 2012 conduit d'une mission d'inspection et de contrôle portant sur les heures des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des masseurs-kinésithérapeutes. la ministre de la Santé et des solidarités Agnès Buzyn, a conscience que certaines modifications qu'il reviendra aux heures de mettre en oeuvre vont impacter évidemment leur fonctionnement habituel mais les objectifs poursuivis ne sont pas discutables et à la confiance dans leur capacité d'adaptation, confiance qui est partagé d'un évidemment pas l'ensemble du gouvernement, ce qui importe désormais ce sont véritablement que les objectifs communs vers lesquels les ordres doivent converger les phases de transition constitue dans ses perspectives des étapes, des étapes que tout le gouvernement s'est attaché à faciliter en émettant des avis favorable à plusieurs mesures d'ajustement proposé lors de la présentation du texte à l'Assemblée nationale.

Il s'agit là en la circonstance d'accompagner et de préparer les acteurs à mettre en oeuvre les nouvelles dispositions prévues dans les meilleures conditions possibles, gage d'une intégration durable et réussie des nouvelles mesures adoptées. De ce fait, nous serons attentifs à ce que les dispositions transitoires qui rejoindra prendre par décret pour mettre en oeuvre ces dispositions soit animé du même esprit, permettant d'accompagner au mieux les ordres dans la datation de ces réformes. Plusieurs des amendements adoptés lors de l'examen du texte par votre commission des affaires sociales, n'entrent pas précisément dans cette perspective, mais au contraire à remettre en cause des dispositions structurelles, c'est la raison pour laquelle le gouvernement ne peut il y a être favorable, l'ordonnance se divise en 3 chapitres qui concernent le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, et enfin les dispositions transitoires et finales le chapitre 1er concernant le code de la santé publique, conforte le contrôle à l'échelon national désordres suivi la politique immobilière de l'ordre certification des comptes combinés au niveau des conseils nationaux, application des principales règles des marchés publics à etc et renforce les notions d'impartialité et d'indépendance, tant pour les conseils que pour les chambres disciplinaires, présidée par un magistrat incompatibilité limite d'âge, durée du mandat condition détermination et publicité des indemnités etc etc. Le chapitre 2 concerts, le code de la sécurité sociale et applique aux sections des assurances sociales, de la Chambre disciplinaire, les conditions d'exercice des conseillers d'État et des magistrats administratifs qui en assure la présidence, et enfin, le chapitre 3 regroupe les dispositions transitoires et finales distingue les articles du code de la santé publique, issue de la présente ordonnance et les feux, entrer en vigueur au lendemain de sa publication au moment de sa publication sur l'ordonnance de mise en cohérence des textes pris en application de la loi de modernisation de notre système de santé quelques éléments, cette ordonnance a été voulue par le législateur au moment du vote de la loi pour permettre la mise en cohérence à droit constant des dispositions existantes connexes avec les dispositions nouvelles introduites par la loi et de supprimer des dispositions devenues obsolètes ou devenues redondantes, c'est une opération qui est synonyme de meilleure lisibilité du droit et de la sécurité juridique, le délai d'habilitation s'étend jusqu'au 26 janvier 2018 certaines coordination et opportune étant d'ores et déjà disponible, elles ont donc c'est l'objet d'une première ordonnance c'est celle-ci que le gouvernement vous demande de bien vouloir ratifier. Il y aura d'ici au 26 janvier 2018 une seconde ordonnance de coordination si il les débats révèlent des besoins de coordination non satisfaits. L'ordonnance de la ratification et demandé conscient de blocs de dispositions le titre 1er article 1er, 2, 3 et 4 modifie les dispositions de code de la santé publique, de la sécurité sociale, de l'éducation et du code général des impôts pour tirer les conséquences de la réintroduction par par la loi du service public hospitalier. La réaffirmation du service public hospitalier a pour intérêt de donner davantage de lisibilité aux patients et aux patientes dans l'offre hospitalière. Le service public hospitalier a en effet été ouvert à l'ensemble des établissements de santé, indépendamment de leur statut. Il repose non plus sur une liste de mission mais sur des obligations de service public qui s'impose aux établissements de santé, faisant le choix du service public hospitalier. Parmi ces obligations figurent notamment l'égalité et la permanence de l'accès aux soins ou encore l'accessibilité financière. L'ordonnance précise notamment l'articulation entre les dispositions sur le service public hospitalier et celles relatives à l'activité libérale des praticiens et des praticiens hospitaliers. Le titre 2 articles, 5, 6, 7 et 8 procède par ailleurs à des adaptations nécessaires dans les domaines plus divers, notamment je vous en lister quelques-uns sur le partage des informations au sein de l'équipe de soins les berges données santé à caractère personnel, la concertation avec les représentants de les représentants des associations d'usagers, le développement personnel continue des professionnels de santé, la fusion des collèges de médecins spécialistes, la détermination de zones géographiques caractérisées par des offres de soins soient surdotées soit sous-dotées et enfin la fusion des comités consultatifs nationaux, des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Monsieur le président, le seul président de la commission des affaires sociales Madame la rapporteur mesdames et sénatrice de messieurs les sénateurs, quel était le détail

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, un très grand nombre d'ordonnances 33 ce jour ont été publiés au titre de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, nous examinons aujourd'hui les projets de loi de ratification de 4 d'entre elles, dont les dispositions sont de nature et de porter extrêmement diverses, 2 de ces textes ont été approuvé sans modification par la commission des affaires sociales, l'ordonnance de mise en cohérence des textes et celle relative à la profession de physicien médical, la Commission a salué la reconnaissance dans la loi de cette profession de santé cette avancée répond à une attente forte des acteurs concernés, il y a une double exigence de sécurité et de qualité des prises en charge, ailleurs, a part ailleurs approuvé la ratification de l'ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé tout en ajustant plusieurs de ses dispositions, certaines mesures vont dans le bon sens en améliorant la transparence interne de ses instances ou en renforçant les exigences d'indépendance et d'impartialité, elles sont de nature à conforter la nécessaire confiance des professionnels de santé à leur égard, toutefois, la Commission s'est interrogé sur la pertinence d'autres évolutions susceptibles de faire peser sur les ordres de lourdes charges de gestion les soumettre à des procédures de marchés publics paraît quelque peu disproportionné, alors que des ordres se sont déjà auto-responsabiliser sur ce sujet, la commission a également estimé inopportune la possibilité nouvelle de remplacement des pharmaciens d'officine, en tout cas, entre guillemets, de circonstance, exceptionnel, alors que la loi santé avait déjà permis une avancée pour tenir compte de situations individuelles. Sur la forme, l'articulation de l'ordonnance que nous nous apprêtons à ratifier et d'une autre publiée 2 mois plus tôt, pose quelques difficultés de lisibilité du droit en outre la décision de ne ratifié qu'un seul de ces textes interrogé. Peut-être pouvez-vous nous éclairer, Madame la Ministre, sur la stratégie du gouvernement concernant le calendrier de ratification des nombreuses ordonnances prises sur le fondement de la loi santé sur le fond, je souhaiterais attirer votre attention, madame la ministre, sur 2 points qui m'ont été relevés au sujet de l'ordonnance de février 2017, le 1er porte sur la limite d'âge de 71 ans révolus applique la candidat aux élections ordinale cette notion a donné lieu à des interprétations divergentes une clarification de votre part permettrait de sécuriser les opérations de renouvellement qui vont s'échelonner dans les mois à venir. Le second point concerne des effets contre-productifs des binômes d'élus visant à favoriser la parité au sein des conseils du no comment entendez-vous prendre en compte les difficultés concrètes constatés par certains ordres à l'occasion de récentes élections je terminerai en l'abordant plus longuement par la plus sensible, des questions, celle de l'accès partiel des ressortissants européens aux professions médicales et paramédicales, porté par l'ordonnance transposant une directive européenne de 2013. Ce sujet certes technique, mérite une attention particulière de notre assemblée. En effet, ces dispositions pourrait avoir des conséquences très importantes sur l'organisation et la cohérence de notre système de santé la mise en place d'un accès partiel sous l'impulsion des instances communautaires, c'est expliquent par les différences de choix des États-membres quant à l'organisation de leur système de santé articulé autour de professions dont les contours ne se recoupent pas nécessairement d'un pays à l'autre, faut-il pour autant au motif d'assurer la liberté d'établissement et la libre prestation de services, des professionnels de santé européens, remettre en cause la cohérence de notre propre organisation des soins, la commission des affaires sociales a estimé que non, elle a, en conséquence, choisi d'abroger les dispositions relatives à l'accès partiel en se fondant sur 4 séries de reconsidération notre commission a en 1er lieu été frappé par le degré d'impréparation entourant la mise en place d'une évolution aussi fondamental à l'heure où nous a demandé de ratifier cette ordonnance, on ne dispose ainsi d'aucun élément d'évaluation sur le nombre de professionnels susceptibles de formuler une demande en France ou sur la nature même des professions qui pourraient être concernés, madame la ministre des solidarités et de la santé, a indiqué qu'une cartographie des professions de santé des États-membres avait été demandé aux instances communautaires me semble cependant que cette demande intervient un peu tard, comment sans connaître les professions, le gouvernement peut-il prétend préparer un texte d'application garantissant la sécurité de l'ensemble des situations, il me semble que l'on avance ici à l'aveugle et si vous me pardonnez l'expression que l'on mettrait la charrue avant les boeufs en autorisant un dispositif dont nous ne connaissons pas la réalité et de la portée concrète en second lieu, cette mesure me semble nature à désorganisé en profondeur l'organisation de notre système de santé qui n'est certes pas parfaite, mais au moins le mérite de garantir généralement la qualité et la sécurité des soins. Il ne s'agit pas ici de faire un procès d'intention professionnels dans d'autres pays, dont je ne remets pas en cause la compétence, c'est la compatibilité de l'accès partiel avec l'organisation et l'efficacité de notre système de santé que j'interroge ici il me semble, ce point de vue que la reconnaissance d'un accès partiel ne pourra qu'aboutir à une fragmentation des professions dont on peine encore à mesurer toutes les conséquences, je me demandais si comment les services hospitaliers pourront fonctionner avec des équipes réunissant des professionnels n'ayant pas tous le même Champ de compétence, comment pourra-t-on contrôler qu'un professionnel exerce en libéral n'outrepasse pas le Champ de ses compétences, je vous avoue également ma perplexité à l'heure où le débat semble plutôt porter sur une élévation de la qualité professionnelle des médicaux et des paramédicaux dans le cadre européen LMD et où l'enjeu majeur paraît plutôt résider dans le développement des coopérations interprofessionnelles dans ce contexte, la création et je mets entre guillemets de sous-profession j'utilise cette expression sans jugement de valeur, ne pourra que renforcer la complexité de notre organisation des soins. Il est ensuite permis de redouter et c'est ma 3ème observation que les problèmes de qualité et de sécurité des soins ne frappe d'abord les patients les moins informés et donc les populations les plus fragiles, on pourrait même craindre sans céder à une trop forte méfiance que ces professionnels soient opportunément recruté par des établissements de santé en pénurie de personnel ou par nos collectivités frappées par la désertification médicale, cela serait de nature à renforcer les inégalités territoriales de santé. Jean vient en dernier lieu aux difficultés pratiques pointées lors de mes auditions d'abord le surcoût potentiel pour la sécurité sociale si des patients se trouvent contraints de consulter 2 professionnels au lieu d'un, compte tenu de la limitation des compétences du 1er ensuite l'effet d'aubaine pour les formats formateurs étrangers notamment, alors que la formation des projets personnels médicaux ces paramédicaux fait déjà l'objet d'un marché très disputé dans certains pays de l'Union européenne, enfin, sur la sécurité réellement garantir aux patients alors que des difficultés importantes sont d'ores et déjà constater dans le cadre de la procédure de reconnaissance automatique s'agissant notamment de la compétence linguistique des professionnels ou de leur niveau réel de formation, nous aurons l'occasion d'évoquer cette question de la maîtrise de la langue lors de la discussion d'amendements déposés par plusieurs de nos collègues, la commission des affaires sociales, je tiens à le souligner, a bien pris la mesure, à la fois des obligations communautaires pesant sur la France de l'analyse juridique du Conseil d'État, des garanties apportées par le gouvernement au dispositif, ainsi que de la menace d'éventuelles sanctions européennes en cas de défaut de transposition, elle ne saurait être taxé d'irresponsabilité sur ce point, il nous a au contraire semblé qu'ils relevaient de notre responsabilité de ne pas faire passer la satisfaction d'une obligation d'autres juridique avant l'intérêt des patients, j'ai d'ailleurs pu observer au cours des auditions que j'ai conduite que l'ensemble de ces observations étaient largement sinon unanimement partagé par les acteurs du monde de la santé, les professionnels de santé se prononce d'une seule voix en faveur du retrait de cette mesure, il est à cet égard révélateur que les arguments invoqués par le gouvernement à l'appui de la ratification de cette ordonnance de porte que sur les obligations communautaires de la France et non sur l'intérêt intrinsèque de la procédure d'accès partiel pour l'évolution de notre système de santé il me paraît dès lors invraisemblable de sacrifier contre la vie de tous les acteurs de la santé, la qualité des soins à des considérations essentiellement juridique, l'Allemagne a quant à elle fait un autre choix de transposition en ouvrant pas l'accès partiel à l'ensemble des professions de santé, même s'il y a si vous l'avez rappelé, elle pourrait se trouver exposés à des sanctions européennes, cela montre qu'une nouvelle négociation est encore possible et même souhaitable et que le gouvernement devrait avant tout oeuvrer à trouver une solution acceptable pour tous au niveau européen. Quelles sont, monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des Affaires sociales, mes chers collègues, les principales observations et conclusions de la commission des affaires sociales sur ces textes qu'elle vous demande d'adopter, je vous remercie de votre attention. Dans la suite de la discussion commune, la parole est à Madame Patricia Schillinger pour le groupe, la République en marche 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission madame la arabe le rapporteur mais, chers collègues, les 3 projets de loi rate de ratification que nous examinons aujourd'hui dans une discussion commune découle de différentes habilitation d'ordonnances contenues dans la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, elles répondent à des objectifs et des enjeux qui leur sont propres, s'agissant du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 12 juin, janvier 2017 relative à la mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé le groupe la République en marche votera sans réserve ce texte adopté sans modification en commission des affaires sociales, les articles 9 de l'ordonnance opère diverses coordinations principalement au sein du code de la santé publique du code de la sécurité sociale du code général des impôts et n'appellent pas de remarque particulière de l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, notre groupe soutient pleinement l'objectif de faire évoluer les compétences des organes désordre concernés de consolider leurs règles de gestion interne et enfin de renforcer l'indépendance et l'impartialité de juridiction ordinale certes la mesure visant à rendre applicable aux conseils nationaux de grands le grand peu les grands principes de marché public va modifier en profondeur leur fonctionnement et l'on comprend que certaines réticences s'expriment pour autant l'objectif poursuivi n'est pas discutable puisqu'il vise à rendre applicable, les principes de liberté d'accès à la commande d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures aussi le groupe la République en marche ne veut soutenir ne peut soutenir la position de la commission qui a supprimé les dispositions en matière de marchés publics, l'approche de l'Assemblée nationale qui a allongé la période de transition jusqu'au 1er janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2019 nous semble préférable car elle permet à la fois de répondre aux recommandations de la Cour des comptes et de laisser aux ordres, le temps nécessaire afin de s'adapter, c'est pourquoi, en l'état du Texas, nous nous abstiendrons sur ce second projet de loi s'agissant enfin du dernier projet de loi ils procèdent à la ratification de 2 ordonnances distinctes du 19 janvier 2017 à l'article 1er la ratification de l'ordonnance relative à la profession de physicien médical et à l'article 2, celle relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles la première consacre la profession de physicien médical en tant que profession de santé défini le cadre général de la profession et l'émission de physiciens, le tout au terme d'un fructueux travail de concertation avec les représentants des physiciens médicaux et des spécialités médicales concernées, cette avancée qui répond à l'un des objectifs du plan de cancer 2014, 2019 permet également de donner une suite constructive aux recommandations du comité national de suivi des mesures nationales pour la radiothérapie après l'accident se renier à et à ce texte contribuera à renforcer la qualité et à améliorer les pratiques dans le domaine de l'utilisation des rayonnements ionisants tout en sécurisant l'exercice de la profession, le groupe la République en marche votera donc l'article 1er du projet de loi qui s'inscrit dans l'amélioration de la qualité des soins du de notre système de santé, je viens pour terminer à l'article 2 et à l'ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, l'ordonnance procède à la transposition dans notre droit de la directive 2013, 55 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, en particulier de 3 dispositions la carte professionnelle européenne l'accès partiel et le mécanisme d'alerte la transposition proposées suscite des inquiétudes des professionnels de santé dans nos travaux en commissions se sont largement fait l'écho, l'inquiétude porte en particulier sur l'accès partiel aux professions de notre système de santé au risque de fragmentation des professionnels de santé, voire de mise en cause de la qualité de la sécurité des soins, Madame la Ministre, vous avez exposé le contexte et les raisons juridiques qui conduisent aujourd'hui le gouvernement a procédé sans plus attendre à cette transposition pour 30 pour l'ensemble des professions de santé sans exemption, même partielle, le groupe la République en marche vous apporte son soutien dans les choix responsable qui est de est le vôtre de ne pas ex exposer la France à une procédure pour défaut de transposition, alors qu'elle a déjà reçu 2 avis motivé de la Commission européenne, rappelons par ailleurs que des garanties existent pour contenir des risques et inquiétude à travers les 3 conditions cumule Tati posés par la directive transposée le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son état d'origine, l'activité pour laquelle pour laquelle il est sollicité un accès partiel les si les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'état d'origine et la profession qui pourrait lui correspondre en France sont importantes, il faudra appliquer des mesures de compression compensation de formation qui reviendront à faire suivre aux demandeurs d'un enfin l'activité en accès partiel doit pouvoir être l'objectif séparé d'autres activités relevant de la profession, correspondante en France c'est l'une des ces 3 conditions n'est pas rempli l'autorisation d'exercice partiel ne pourra être délivré, nous serons donc partie Kelderman attentifs aux mesures réglementaires qui seront adoptées sur la base de cette ordonnance et leur mise en oeuvre concrète, compte tenu des amendements adoptés en commission qui à notre avis, expose la France à des poursuites, nous nous abstiendrons sur le vote de l'article 2 du projet de loi, je vous remercie. La parole est ta Monsieur Dominique Vatrin pour le groupe communiste républicain et citoyen et écologiste. Oui, tout d'abord une pensée pour notre collègue Laurence Cohen, touché par un deuil familial, monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le Sénat est appelé à ratifier 4 ordonnances prévues par la loi de modernisation de la santé avec les autres membres du groupe CRC, nous avions voté contre cette loi dont nous ne partageons pas la philosophie générale serait d'ailleurs intéressant d'en faire un bilan, notamment sur l'une de ses principales dispositions, savoir des groupements hospitaliers de territoire au lendemain d'une journée de grève dans la fonction publique qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants je souhaiterais au préalable, rendre hommage aux personnels de la fonction publique hospitalière, ces hommes et ces femmes se battent au quotidien pour soigner les patients dans des conditions de travail de plus en plus dégradé, avec des rémunérations bien en deçà de leurs qualifications et des horaires à rallonge, l'hôpital est aujourd'hui au bord de la crise de nerfs, avec le non-remplacement des départs en retraite causées par des années d'austérité financière imposée par les gouvernements successifs, notre groupe est le seul à s'être opposé de manière constante ainsi régression car nous avons toujours estimé que l'humain devait primer sur la finance et non l'inverse de la même manière, nous nous sommes toujours opposés à l'utilisation des ordonnances qui retire aux parlementaires leur pouvoir de législateur concernant l'ordonnance sur l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement désordres des professions de santé, je rappelle l'opposition de principe de notre groupe aux ordres professionnels se sont en effet des organisations corporatistes défendant des intérêts particuliers d'une catégorie professionnelle contrairement aux syndicats qui défendent les intérêts professionnels de l'ensemble des travailleuses et travailleurs sans distinction, par ailleurs, les évolutions proposées ici ne règle pas les véritables dysfonctionnements constatés des professionnels dépourvus en réalité de système démocratique et de véritables instances représentatives du personnel et c'est pourquoi nous voterons contre cette ordonnance concernant l'ordonnance relative à la mise en cohérence des textes comme les mois permettez-moi d'illustrer nos critiques sur le recours abusif aux ordonnances lors de l'examen de la loi dite de modernisation de la santé, l'article 225 prévoyez, je cite, d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente il y a abrogé des dispositions devenues sans objet, une phrase tellement vague à laquelle il semble difficile de s'opposer, pourtant derrière cette formule, le gouvernement de l'époque a essayé de mettre un terme à un imbroglio juridique, il était en effet interdit aux professionnels du secteur privé, d'exercer une activité libérale à l'hôpital public, tandis que les praticiens hospitaliers du public pouvait continuer à pratiquer des dépassements d'honoraires l'ordonnance explicite donc l'articulation entre le principe de l'interdiction des dépassements d'honoraires au sein du service public hospitalier et le maintien d'une dérogation possible dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein, alors que près d'un quart des Françaises et des Français renoncent ou reportent leurs soins dans l'année, principalement en raison des dépassements d'honoraires, nous proposons de supprimer la possibilité pour les professionnels de santé exerçant dans les établissements cru Blick de pratiquer des dépassements d'honoraires, enfin, concernant le dernier projet de loi de ratification de leur donnant s'relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et celle relative à la profession de physicien médical, nous sommes satisfaits, la suppression par la commission de l'accès partiel aux aux activités médicales ou paramédicales, mais nous continuons à refuser la libéralisation des professions réglementées imposée par l'Union européenne dans une logique de nivellement par le bas et de remise en cause des qualifications, nous demandons aussi de reconnaître la maîtrise de la langue comme faisant partie du Champ des compétences, des orthophonistes, afin de garantir aux patients souffrant de trouble du langage, des soins de qualité, il est indispensable que les orthophonistes maîtrisent eux-mêmes la langue française, c'est le sens de l'amendement que nous avons déposée, enfin la création de la profession de physicien médical comme une profession de santé à part entière, est une bonne nouvelle, d'autant que leur nombre et l'encore largement insuffisant au regard des besoins de notre pays et pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce dernier projet de loi de ratification. La parole est maintenant à monsieur Van Renberg pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la ministre, monsieur le président de la commission madame le rapporteur mais, chers collègues, nous débutons donc cette session parlementaire avec 3 projets de loi de ratification d'ordonnances qui sous des aspects très techniques, aborde des sujets particulièrement important, tiens tout d'abord à remercier notre rapporteur Corinne Imbert pour son excellent travail très complet et documenté et tout cela au coeur de l'été, je ne reviendrai pas sur le 1er projet de loi qui ratifie l'ordonnance de mise en cohérence des textes au regard de la loi santé qui n'appelle pas de commentaire particulier. Ce n'est pas le cas du second projet de loi, en tout cas en ce qui concerne l'ordonnance ouvrant l'accès partiel aux professions médicales et paramédicales. Je partage comme l'ensemble de mes collègues du groupe de l'Union centriste, les réticences de Madame Imbert sur cette disposition, elle fait en effet peser des risques inconsidérés sur l'organisation de notre système de santé d'une part, mais surtout sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Sion, pardon, des règles en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'Union européenne participe à son renforcement, cela est indéniable, les professions de santé ne doivent pas il y a échappé, elles doivent en revanche faire l'objet d'une attention particulière, comme du reste toute réglementation les concernant, pour des raisons dessus de sécurité des patients que je viens d'évoquer, comme l'a rappelé Corinne Imbert plusieurs professions médicales bénéficient déjà d'une reconnaissance automatique leur permettant d'exercer dans un pays différent de celui dans lequel ils ont été formés, c'est le cas des médecins, infirmiers, dentistes, sages-femmes et pharmaciens dont les exigences minimales en matière de formation ont été harmonisées en au niveau communautaire, cette mesure est essentielle pour notre propre système de santé dont le fonctionnement est assuré en partie par ces professionnels de santé venus d'autres pays européens, elle permet notamment de participer à l'accès aux soins et de lutter contre les déserts médicaux. Mais je suis en revanche nettement moins favorable à l'accès partiel ouvert par cette ordonnance et la directive qu'elle transpose au professionnels ne pouvant bénéficier de la procédure de reconnaissance automatique. Je ne reviendrai pas sur le fonctionnement de ce dispositif qui a été parfaitement décrit préalablement. Mais le principe qui est dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne se comprend en soi mais comme je le disais, ne peut être adaptée de manière absolue aux professions médicales en dépit de ses difficultés, notre système de santé est organisé et solide, il ne peut souffrir de l'arrivée de professionnels en partie et seulement en partie compétents, sans que cela ne présente des risques pour la sécurité des patients, vous en conviendrez, à l'heure où on parle d'une amélioration des parcours de santé de pertinence des soins, peut-on envisager d'ajouter des difficultés supplémentaires. Je crois pas cela opportun, nous avons effectivement des besoins en terme d'accès aux soins afin de lutter contre les déserts médicaux, mais l'accès partiel pourrait être envisagée par certains comme une solution. Et je pense quant à moi qu'il faut des médecins, des infirmières, des dentistes pleinement formée. Et compétents. Et donc nous nous opposerons avec le reste de mon groupe à cette disposition en votant la version de la commission des affaires sociales, j'ai d'ailleurs noté dans votre rapport Madame le rapporteur madame Himbert que l'Allemagne avait refusé. Cet accès partiel qui nous expose d'ailleurs à des sanctions de l'Union européenne ne pourrait-on envisager, madame la ministre, la question s'adresse à vous et au gouvernement d'engager avec les Allemands. Une procédure commune de modification de la directive européenne pour tenir compte de tous ces remarques qui viennent de tous les bons. Le dernier projet de loi concerne la ratification d'une ordonnance sur les ordres des professions de santé, me semble-t-il, que les règles applicables à ces structures soient quelque peu revu afin d'gare à garantir la fiabilité. à ce titre, les recommandations du Conseil d'État de l'IGAS et de la Cour des comptes sont bienvenues et nous le retrouvons dans ce texte, elle concerne la transparence, naturellement, mais aussi les exigences d'indépendance et d'impartialité des instances disciplinaires ces acteurs sont utiles dans la définition et l'organisation de notre système de santé, il est donc souhaitable et normal qu'il soit soumis à des règles communes garantissant leur bon fonctionnement, nous votons donc ce 3ème projet de loi telle qu'amendée par la commission des affaires sociales. Voilà le gouvernement sur le fond n'est pas responsable des taxes qui nous sont présentés aujourd'hui ses premières réformes, on le sait, sont à venir en matière de santé nous seront proposées, vraisemblablement à l'occasion du prochain prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le groupe de l'Union centriste fera preuve à cette occasion de la même analyse qui préside à notre prise de position sur ces 3 projets de loi, c'est-à-dire maintenir la cohérence de notre système de santé en corriger les imperfections évidemment sans l'alourdir de règles inutilement complexes ou au contraire l'alléger imprudemment donc dans l'immédiat nous voterons donc ces 3 projets de loi telle qu'amendée par la commission des affaires sociales, je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Yves Deligny pour le groupe socialiste et républicain.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission, même le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur 3 projets de loi de ratification d'ordonnances rédigées en application de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 loi votée à l'initiative de la précédente ministre de la Santé, Marisol Touraine, que nous avions soutenue dans sa démarche, notre attitude, je parle évidemment de mon groupe aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de ce positionnement, l'ordonnance de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé permet d'harmoniser à droit constant, les dispositions en vigueur, elle répond aux exigences élémentaires de sécurité juridique, j'insiste sur le titre 1er qui modifie les dispositions de 4 codes pour tenir compte de la réintroduction par la loi du service public hospitalier la référence aux missions de service public, instituée par la loi dite HPST de juillet 2009 et supprimer des obligations de service public s'impose maintenant aux établissements de santé ayant fait le choix du service public hospitalier, il en résultera davantage davantage de visibilité pour les patients, dont l'offre hospitalière l'ordonnance relative à l'adaptation des dispositions relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, renforce l'indépendance et l'impartialité des juridiction ordinale fait évoluer les compétences des organes désordres et permet l'application par leurs conseils nationaux de la législation relative aux marchés publics, si certaines des modifications qu'il reviendra aux ordres de mettre en oeuvre affecteront leur fonctionnement habituel, les objectifs visés ne me semble pas l'ordonnance relative à la profession de physicien médical qui concerne quelque 650 personnes reconnaît la profession de physicien médical comme une profession de santé malgré le niveau de qualification très élevée qu'elle requiert cette profession n'avait toujours pas reconnue comme telle, répondant à l'un des objectifs du plan cancer 2014, 2019 la reconnaissance du métier de physicien médical contribuera non seulement à sécuriser à sécuriser les pratiques mais aussi à reconnaître son apport incontestable à l'amélioration de la qualité des soins, c'est en donnant, je veux souligner, fait suite à un important travail de concertation menée depuis juin 2016 avec les représentants des physiciens médicaux et des spécialités médicales concernées, j'en viens alors donnant s'relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, elle transpose en droit interne 3 dispositifs mis en place par une directive européenne de 2013 la carte professionnelle européenne le mécanisme d'alerte et l'accès partiel, les 2 premières constitue une avancée en matière de coopération entre États membres sur lesquels il n'est pas nécessaire de s'appesantir pardon de l'exercice partiel sur lequel reviendra précisément avec tout le talent qu'on lui connaît tout à l'heure, mon collègue Jean-Louis Touraine soulève plus d'interrogations ou d'inquiétude certes, nos voisins allemands n'ont pas transposé la directive allait être prêt, mais vous avez affirmé, Madame la Ministre qu'exemptés toutes au parti des professions de santé du Champ d'application n'était ni souhaitable ni concevable au regard du droit et de la jurisprudence européenne, je veux rappeler d'abord que l'accès partiel ne serait pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leur qualification professionnelle, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, difficile de penser que la mise en place du dispositif déstabiliserait l'ensemble de notre système de santé je veux ensuite souligné les 3 conditions générique par la directive et devant entrer autre pour mettre en oeuvre un processus de dépôt et d'examen de dossiers en vue d'obtenir une autorisation d'exercice partiel, il sera bien entendu nécessaire de revenir sur ce sujet qui a été supprimée du texte par la commission des affaires sociales du Sénat par la majorité du Sénat et qui, rappelons-le, une fois de plus, aurait dû être transposée dans le droit français au plus tard le 18 janvier 2016, je vous remercie. La parole est à Monsieur Daniel Chassain du groupe républiques et et Territoires les indépendants. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le président de la commission Madame le rapporteur mais, chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter notre collègue Colin Corinne amer pour son rapport clair et documenté sur ces 3 projets de loi le 1er ratifie une ordonnance procédant à divers corps

dans le milieu hospitalier dans les centres de lutte contre le cancer, leur rôle dans la sécurité de 1er plan, nous nous souvenons des problèmes graves survenus à Epinal et à Toulouse, il s'agit donc de renforcer les dispositions relatives aux physiciens médicaux et d'aboutir à une meilleure définition de leur rôle et de leur mission est de clarifier leur responsabilité au niveau d'une équipe pluridisciplinaire, l'ordonnance intègre la profession dans le code de la santé publique, avec une définition et prévoit les conditions d'exercice, nous sommes favorables à cette ordonnance la 2ème ordonnance qui a été retiré par la commission et celle de l'accès partiel aux professions médicales et paramédicales, donc je souhaitais malgré tout en dire quelques mots, car le problème persiste vis-à-vis de l'Europe, et bien sûr pourrait pas réglé dans les pays de l'UE, il y a une procédure de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles permettent à certains professionnels de l'exercer dans un autre pays, la liste des diplômes des diplômés, fixé par la directive de 2005, ça les médecins, ça a été dit, dentistes, sage-femmes, pharmaciens, les infirmiers de soins généraux, mais pour les professionnels de bénéficiant pas de cette procédure automatique, la cour a estimé que l'État d'accueil devait les autorisés à exercer en limitant les tâches pour lesquelles ils sont compétents, il s'agit de nouveaux dispositifs d'accès partiel

avec des sanctions européennes possible en cas de non disposition puisque ça fait maintenant près de 3 ans de 2 ans qu'il y a un retard il y a des professions où l'accès est possible, vous l'avez cité Madame le rapporteur comme le pédicure-podologue il est indiqué aussi dans ce projet de loi que certaines mesures hé bien bon pour moi dans le bon sens pour sécuriser les patients vis-à-vis des professionnels, la mise en place d'une carte professionnelle, les conditions pour exercer un accès partiel dont acte pleine qualification dans le pays, maîtrise de la langue examen au cas par cas des demandes auprès de l'État a dit de Delors, c'est quand même qu'on a dit consultatif refus pour des raisons d'intérêt général, une commission de spécialistes qui examinerait le dossier, tout comme l'article IV effectivement s'il y a beaucoup de différences entre l'activité professionnelle de l'état d'origine et l'état d'accueil, on aura une formation mais ça aura une coup on reconnaît, Madame la Ministre, que ce sont des sécurités indéniable mais nous ne disposons pas d'éléments d'évaluation sur le nombre de professionnels, ni sur la nature exacte des professions concernées de plus l'accès partiel va aboutir à une fragmentation des professions et ce sera vraiment difficile pour les patients, alors bien sûr, je rappelle à nouveau que les médecins, infirmiers de soins généraux, dentistes, sages-femmes ne sont pas concernés par cette ordonnance, mais le rapport indique que le masseur balnéo thérapeute et kinésithérapeutes sont assimilé les faire moins l'effet des infirmiers de soins généraux ne sont pas concernés, mais la fermer spécialiste alors certains professionnels considèrent même que cette loi pourrait constituer une dérogation aux professions concernées par la reconnaissance de 2005, qu'en est-il exactement, Madame le ministre, alors qu'il y a des difficultés dans la procédure de 2005, liée à la langue et quelquefois au au niveau réel de formation et d'expérience, nous souhaitons davantage d'informations sur le projet de loi concernant cette l'accès partiel aux professions médicales et paramédicales des professions de santé et nous-mêmes souhaitons savoir quelle profession exactement envisagé cours, nous connaissons problème juridique qui aurait dû être évoqué il y a longtemps mais ne pourrait-on pas avoir une prorogation de cette date pour avoir plus d'informations et ainsi identifier clairement les professions de santé, je pense que, avant tout ça, il est nécessaire que les patients et les professionnels et davantage de précisions, le 3ème projet de loi prévoit de ratifier l'ordonnance du 27 avril relative au fonctionnement des ordres des professions de santé, alors elle a pour objet d'appliquer aux conseils nationaux des procédures d'adoption des marchés publics de renforcer l'échelon national pour règlement intérieur une publication de rapports d'activité, la certification des comptes incompatibilité entre les fonctions ordinale et syndicats, l'Assemblée nationale a complété l'article 2 concernant les indemnités du président, l'article 3, coordination et là j'mis des magistrats article 4 des compatibilité s'appliqueront renouvellement des instances, l'article 5. Report en 2020, au lieu de 2019, ce projet de loi pour nous ne pose pas de problème, en conclusion, bien sûr, nous sommes favorables au projet de loi de coordination, le 2ème projet de loi très favorable pour la position de physiciens en ce qui concerne l'accès partiel aux professions médicales et paramédicales, il a été retiré par la commission 3ème projet de loi, nous sommes favorables au fonctionnement des ordres professionnels de santé maire. La parole est à monsieur Guillaumard, Neil du Rassemblement démocratique et social européen pour 6 minutes.

Monsieur le Président, Madame la ministre Madame la rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs, mes chers collègues. Ce projet de loi de ratification que nous examinons aujourd'hui concerne 4 ordonnances prises en application de la loi de modernisation de notre système de santé promulguée en janvier 2016, comme l'a si bien exposé Madame la rapporteure Corinne Imbert que je félicite pour la clarté de son rapport, malgré la complexité en la matière, la première ordonnance relative à la mise en cohérence des textes ne pose aucun souci particulier inutile donc de commenter outre mesure la seconde ordonnance relative à la profession de physicien médical est particulièrement intéressante. En nous plongeant dans l'examen de ces projets de loi, nous sommes nombreux à avoir découvert cette profession qui ne compte aujourd'hui qu'environ 650 praticiens. Les substances radioactives utilisées à des fins thérapeutiques sont indiscutablement des outils à manier avec précaution, et ce n'est pas anodin de reconnaître les compétences particulières des physiciens médicaux en la matière car il contribue à la protection aussi des manipulateurs et surtout garantir l'intégrité des patients, cela devrait permettre d'éviter ainsi les accidents que nous avons eu à déplorer, par le passé, en raison de sur Exposition le but de cette ordonnance, qui fait l'objet d'un consensus dans l'univers médical et de clarifier les compétences du physicien médical et de définir son cadre juridique d'exercice il n'appelle donc pas non plus de commentaire particulier de ainsi, comme le 1er texte le groupe RDSE votera en faveur de son adoption, j'en viens maintenant au coeur du débat avec cette ordonnance, qui concentre les discussions l'accès partiel à certaines activités médicales et paramédicales, j'entends les arguments de ceux qui y sont défavorables, comme vous Madame la rapporteur je veux rappeler brièvement quelques l'impréparation de notre pays à sa mise en place ne connaissant ni exactement le nombre de professionnels qui pourrait en faire une demande ni le type d'activités concernés les conséquences sur notre système de santé seront-elles de nature à bouleverser fondamentalement l'organisation des soins, quelles garanties quant à la qualité des soins fournis et enfin le risque d'accroître encore plus l'inégalité de la qualité des soins, notamment dans les territoires où les structures sont déjà les plus déficitaires en professionnel de santé ou les plus en difficulté. Ses arguments sont ainsi posées, nous conduit à nous interroger, certes, mais au fond il s'articule autour d'une même question est-ce que cette réforme ne va pas se faire au détriment du système de santé de soins et de la complexification de son organisation, nous considérons effectivement, Madame la Ministre, que ces aspects de la problématique que nous étudions aujourd'hui ne sont pas tous s'éclaircit, pourtant, nous ne partons pas avec un a priori négatif sur ce texte, puisque si nous avons écouté les arguments de ceux qui montent ce monde sceptique, voire même pessimiste, nous entendons également les arguments de ceux qui sont en faveur de l'adoption du texte, comme cela a été rappelé, ce projet de loi transpose une directive communautaire que nous aurions dû intégrer dans notre droit national au plus tard en janvier 2000, c'est la première remarque, je formule, c'est qu'on ne peut pas jouer un rôle moteur dans l'Union européenne est fortement contribué à en fixer les règles de fonctionnement sans se les appliquer. Nous avons déjà plus d'un an et demi de retard et c'est vrai, ce n'est pas acceptable la se rendre le Maroc et je l'affirme avec force et sans ambiguïté. Ce que nous avons besoin de l'Europe. Et nous devons, comme les autres États-membres suivent les règles mais selon nos avons besoin c'est d'une Europe qui simplifie qui harmonise qui protège et qui aligne vers le haut les exigences en terme de qualification d'encadrement et de compétences requises, nous ne voulons surtout pas d'une Europe qui nivelle vers le bas le texte répond simplement en partie à cette crainte en prévoyant bien entendu la possibilité de fragmenter les compétences pour en autoriser certaines ayant refusé mais mais cette réponse partielle n'est pas suffisante pour leur dire qu'il sera extrêmement vigilant aux explications que vous fournissez madame la ministre, dans réponse aux interrogations de madame la rapporteure et des autres collègues afin d'en déterminer son vote quant à cette ordonnance en son âme et conscience, enfin, la dernière ordonnance relative au fonctionnement des hommes, des professionnels de santé pour nous nécessaire en ce qu'elle a même la transparence, l'indépendance et l'impartialité des conseils nationaux, je sais que la mise en place des procédures induite par la transparence comme les procédure des marchés publics sont lourds et engendre des surcoûts, mais elles sont indispensables à nos yeux, je note d'ailleurs que l'Assemblée nationale a compléter le projet de loi de plusieurs articles notamment un article 5 juin que l'entrée en vigueur de ces dispositions de 2019 à 2020 pour justement justement laisser à ses ordres, la possibilité de mieux se préparer à la mise en place de ces réformes, Il n'est pas envisageable pour le groupe RDSE de revenir en arrière et de supprimer ces mesures qui tendent vers davantage de transparence, ce que souhaite, très clairement, la majorité de nos concitoyens et ce dans tous les domaines de la vie publique. La parole est à madame Catherine Deroche pour le groupe, les républicains. Pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission des affaires sociales Madame le rapporteur mais, chers collègues, ces 3 projets de loi propose la ratification de 4 ordonnances qui résulte de la loi de modernisation de notre système de santé, je rappelle que nous avions protester contre le nombre inhabituel d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance lors de l'examen de cette loi en effet des articles visait plus d'une centaine d'habilitation dans des domaines très variés, dans la mesure où plusieurs de ces sujets ne présentait pas un caractère purement technique, la majorité sénatoriale avait fait le choix d'en supprimer une grande partie et nous avait semblé indispensable que le Parlement puisse les examiner dans le cadre classique de la procédure législative, il s'agissait notamment des conditions de création et d'organisation des centres de santé et des maisons de santé de l'organisation de la transfusion sanguine de l'accès aux soins de 1er recours du droit applicable aux recherches biomédicales des règles relatives aux ordres des professions de santé, dont nous avons à débattre aujourd'hui tous ces sujets aussi divers qu'ils soient méritait à nous sur un vrai débat au sein des assemblées parlementaires. J'en viens au projet de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi modernisation de notre système de santé la coordination portent notamment sur la suppression de la référence de missions de service public, instauré par la loi hôpital, patience, Santé et Territoires de juillet 2000, nous n'étions pas opposés à la mise en place du service public hospitalier mais nous l'avions complété par le maintien de la possibilité donnée aux établissements privés d'exercer des missions de service public à tarif opposable l'Assemblée nationale avait rétabli sans surprise leur exclusion totale à nos yeux injustifiée d'autant plus injustifiée que cette ordonnance rétablit pour les établissements publics, la possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires pour les praticiens à plein temps, c'est une rupture d'égalité entre des établissements qui pourront être labellisés, secteur public malgré la possibilité d'avoir recours aux dépassements d'honoraires pour leur praticien et ceux qui ne pourront pas nous sommes très attachés à la mixité de notre modèle hospitalier, il existe des complémentarités indéniable entre les établissements publics et privés, malheureusement, pendant ces 5 dernières années, les mesures prises n'ont pas créé les conditions de cette complémentarité, bien au contraire et à vouloir opposer les 2 secteurs, ce sont les patients qui sont pénalisés, nous espérons que cette logique sera abandonnée dans les mois qui viennent, pour le reste du contenu de cette ordonnance, même si nous continuons à le regretter pour certains points, la loi a été adoptée et la mise en cohérence ne peuvent qu'être adopté, s'agissant du projet de loi ratifiant l'ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé, force est de constater que la rédaction de cette ordonnance fait sans concertation avec les professionnels concernés, notre colère et notre collègue Corinne Imbert dans son rapport, nous reconnaissons que cette situation n'est pas de votre fait, Madame la Ministre, mais vous auriez pu envisager la ratification de ces ordonnances sont les synthés, en effet, nous devons nous prononcer sur l'une des 2 ordonnances publiées cette année, pourquoi n'avons pas, n'avons-nous pas à nous prononcer sur les 2, il est surprenant de proposer l'une, 2 ordonnances ratification, alors qu'il s'agit d'une réforme globale, comme le souligne notre rapporteur, je la cite l'articulation entre les 2 textes complexe puisque leur contenu sans cheveux, être sur plusieurs points, le travail du Parlement ne gagne pas en intelligibilité et pire encore, les professionnels de cet ordre. Concernés n'ont pas de lisibilité sur les intentions du gouvernement notre rapporteur s'était attaché à compléter le texte déjà modifié par nos collègues députés afin d'éviter de faire peser des charges excessives sur le fonctionnement et l'organisation désordres nous soutiendrons sans réserve ces modifications, enfin le 3ème projet de loi de rectification aborde des sujets totalement distincts à travers 2 articles, le 1er article relatif à la reconnaissance de la profession de physicien médical comme profession de santé, il s'agit de mieux définir leurs responsabilités dans la prise en charge du patient au sein d'équipes de soins et de reconnaître leur rôle dans la qualité et la sécurité de cette prise en charge, il est utile de souligner que cette mesure est formulée dans le plan cancer 2014, 2000 19 et dans les recommandations énoncées par le comité national de suivi des mesures nationales pour la radiothérapie après les incidents d'Epinal et de Toulouse, ces évolutions étant pleinement soutenue par les professionnels concernés, nous ne pouvons que souscrire à l'article 1er de ce projet de loi, le second article a pour objet la ratification de l'ordonnance qui assure la transposition en droit français la directive 2013, 55 du parlement et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005 36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui introduit notamment la reconnaissance de l'accès partiel aux professions médicales et paramédicales, nous abordons le sujet le plus sensible, sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui nous ne remettons pas en cause la totalité de cette ordonnance nous approuvons par exemple la mise en place d'une carte professionnelle européenne ou encore l'instauration d'un mécanisme d'alerte à l'échelle communautaire dont l'objectif est de garantir la sécurité des patients, en revanche, nous n'approuvons pas l'application d'un accès partiel qui permettre aux professionnels de santé européens qualifiés dans leur pays d'origine, d'exercer en France, sous certaines conditions et seulement pour une partie du Champ d'exercice s'il existe des différences importantes entre leur pays et la France, la mise en place d'un thème mécanisme ne satisfait pas, pour plusieurs raisons, nous constatons un manque d'évolution du dispositif quels métiers seront concernées, quel nombre de professionnels et susceptibles de venir dans notre pays : quelles conséquences sur l'organisation de notre système de soins, toutes ces questions sont sans réponse et nous amène à penser que nous allons ouvrir la voie à une déqualification des professionnels de santé à la mise en place d'un service de santé locaux au final nous pensons qu'il existe un risque majeur pour l'organisation de notre système de santé et de toute évidence, pour la qualité des soins aux patients, par ailleurs, nous ne pouvons pas nous contenter d'un argument juridique sur cette question, la sécurité des patients doit être notre seule priorité, comme cela est évoqué par d'autres collègues, nous vous demandons, Madame la ministre, vous retourner vers l'Union européenne et de négocier, nous ne pourrons pas mettre en place un système alors que nos plus proches voisins européens ont fait un choix différent, je fais référence à l'Allemagne, qui interdit l'accès partiel souffre exception le texte de la directive prévoit lui-même, je le cite, que toute États-membres peut refuser l'accès partiel aux professions de santé, dès lors qu'elles ont des implications de santé publique ou de sécurité des patients sur proposition de notre collègue rapporteur de la commission des affaires sociales a supprimé les dispositions introduisent un accès partiel aux professions de santé au regard des risques pesant sur la cohérence, la qualité et la sécurité de notre système de soins, nous voterons naturellement ce projet de loi telle que modifiée, je vous remercie. la parole est à monsieur Jean-Louis Touraine du groupe socialiste et républicain pour 5 minutes.

minutes. Le président. Madame la ministre, chers collègues, ainsi que l'indiquait Yves de Didier il y a quelques instants, je m'attacherai uniquement dans cette discussion générale a évoqué la partie de l'ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des étrangers communautaires dans le domaine de la santé. Nous avons à ratifier ou non. Une ordonnance de transcription dans notre droit d'une directive européenne. Son caractère communal Touaregs ne saurait pour autant nous priver du droit d'en débattre. Et de nous opposer sur tout ou partie de son contenu, de l'or. Que nous apparaissent des raisons essentielles de le faire. Mais il y en a-t-il. Quelle est la vraie question. 2 remarques préalables me paraissent devoir t'être exprimé. La directive européenne date de 2013 elle modifiait une directrice de, de, d'une directive de 2005, elle est entrée en vigueur en 2014 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoyait la transcription par une ordonnance, ce qui à l'heure de déplaire à bon droit, souvent aux parlementaires que nous sommes. Elle aurait dû figurer dans l'autre droit depuis le 18 janvier 2016, nous devons donc trop tardé, la finalité même de la construction d'un espace européen et d'un d'un espace européen de permettent la libre circulation des hommes, des professionnels des entreprises, des biens et la liberté d'installation. Sommet des obstacles injustifiés reviendrait à compter, à contester une construction bien lente et difficile. Mais qui nous est cher. Ainsi dans l'ordonnance, ce qui nous intéresse aujourd'hui rien normalement ne devrait soulever d'opposition puisqu'il s'agit d'autoriser l'exercice de professions médicales et paramédicales par des ressortissants de l'Union, sous réserve de vérification des tirs formation ses compétences. Ainsi s'applique sans difficulté le droit d'exercer en France pour les personnes ayant obtenu dans leur pays, la qualification d'infirmiers, de sages-femmes de médecins de dentistes ou encore de pharmacien. Elle bénéficie d'un régime de reconnaissance automatique des diplômes puisque les exigences minimales de formation ont été harmonisé au niveau communautaire. Selon les termes du rapport au demeurant excellent, vous avez écrit remarquable mais Le vent ne se lève alors que lorsqu'il s'agit de l'accès partiel à l'exercice d'une profession médicale et surtout paramédical et alors un certain nombre d'objections parfois déconcertante paré de la toutes les vertus sont alors égrené s'apparentant s'apparentant à une instruction uniquement à charge. Le manque de formation. Des professionnels concernés, c'est le 1er argument objection contradictoire quand dans la même présentation, on affirme que l'exigence et la vérification des qualifications constitue l'une des conditions sine économe de l'autorisation. 2ème argument laisse entendre que la frontière entre les pratiques seraient difficiles à déterminer que les débordements pourraient être monnaie courante pourrait etc conditionnel, pourtant il est parfaitement préciser que l'autorisation ne peut intéresser que des activités objectivement c'est Une 3ème garantie forte est apportée l'examen. Au cas par cas permettra, toujours selon le rapport de discerner ce qui peut, le cas échéant, porter atteinte à l'intérêt général en matière de santé publique, on conviendra donc la directive avec son caractère peu contraignant donc inquiétant laisse à chaque pays un large pouvoir d'appréciation, cela vaut-il. Par un éventuel et hop inopportun, refus de la ratification d'encourir des sanctions de l'Union européenne et surtout. De donner le mauvais exemple. Aussi l'idée que nous nous faisons d'une Europe ouverte à la libre circulation des hommes et des biens. Alors que des garanties fortes nous sont apportées nous hein, tout cela nous invite à suivre la proposition du gouvernement, en application de la directive et de la loi de modernisation du système de santé. Sauf à imaginer ce que je ne fais pas. à imaginer des réflexes corporatistes de défense qui serait qui Sierre et mal à notre assemblée, le texte qui nous est présenté doit. Je le crois, le texte du gouvernement devrait être approuvée. Et celui de la Commission. Rejeté. Au cours de la guerre froide. Les Américains dépenser des sommes astronomiques en enseignement pour savoir ce que préparaient les soviétiques. Et se sont aperçus qu'il suffisait d'écouter ce qu'ils disaient pour savoir ce qu'il préparait ce qu'il redoutait. Et c'est ainsi que je et Zaria ainsi les intentions des Soviétiques, hé bien je vous avez largement entendu. C'est. Est-ce que Madame la ministre de prendre la parole, hé bien, prenez la parole.

s'agissant en 1er lieu du calendrier de ratification des ordonnances de la loi de modernisation de notre système de santé, je peux comprendre l'incompréhension sur la dissociation des 2 ordonnances relatives aux ordres, il s'avère que l'ordonnance qui est soumise à votre ratification a notamment pour objectif de faire évoluer les compétences des organes désordres, de permettre l'application aux conseils nationaux désordre de l'ordonnance numéro 2015 899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et de réviser la composition de leurs instances disciplinaires intégrant un certain nombre de recommandations issues du Conseil d'État uniquement ceux qui sont de juridiction administrative et la Cour des comptes, modifiant des dispositions relatives au fonctionnement ordres auxquels ceux-ci peuvent se montrer attaché et élaborer dans un délai contraint par la durée de l'habilitation cette ordonnance a suscité de leur part des réactions et contestation y compris contentieuses aussi face à la charge de travail prévisible des assemblées en début de mandature, le secrétariat général du gouvernement, a privilégié la ratification rapide de cette ordonnance s'agissant par ailleurs de la limite d'âge de 71 ans révolus applicables aux candidates et aux candidats aux élections ordinale, vous m'avez demandé une clarification Oral sur l'interprétation qui est qu'ne donner à cette limite d'âge, compte tenu des différentes interprétations qui ont effectivement été donnée à l'adjectif révolu, il n'apparaît qu'une clarification Oral ne peut suffire à sécuriser les futurs opérations l'étoile désordres qui intégreront la nouvelle d'âge donc cette clarification sera apportée après l'analyse juridique définitive du Conseil d'État, interrogé sur ce sujet et nous ne manquerons pas de la communiquer aux ordres, dès lors qu'elle aura été porté à notre connaissance, s'agissant enfin des binômes d'élus constitué pour favoriser la parité, cette mesure est principalement issus de l'ordonnance numéro 2015 949 du 31 juillet 2015 relatives à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels historiquement et traditionnellement, comme beaucoup d'assemblées élues, les conseils des ordres médicaux et paramédicaux, élus au scrutin uninominal sont demeurés à l'exception d'un n'ordre au coeur de métier très spécifique, c'est-à-dire les sages-femmes sont demeurés à domination très largement masculine ainsi, alors même que les professions de santé, elle même se féminiser les femmes ne constituait qu'une minorité dans leurs instances représentatives afin de garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités dans les ors des professions de santé, le législateur a opté pour le scrutin du nominal, chaque candidat aux ordres devra se présenter en binôme, c'est-à-dire conjointement à un candidat ou une candidate de l'autre sexe, il n'a pas été pour cela nécessaire de doubler le nombre de représentants mais d'aménager la composition de chaque conseil, ce n'est pas utopique cette réforme étendue aux élections des arts, des professions de santé les, dans la continuité d'occasion historique qui nous a été donnée de montrer qu'il est possible de concilier le scrutin majoritaire et la parité que nous nous devons de considérer comme une avancée de la représentativité et de la démocratie, si cette avancée est une première mise en oeuvre cette année pour les uns, professionnels, elle pourra nécessiter après les élections, une évaluation du dispositif et peut-être quelques aménagements techniques, à la marge pour éviter des effets contre-productifs, comme il a pu être constaté par exemple chez les masseurs-kinésithérapeutes salariés ou des femmes, des non à trouver des binômes homme-n'avait pas pu se présenter, il n'est pas envisageable, ni pour le ministère de la Santé, ni donne évidemment pour moi-même, que les autres professionnels de santé connaissent une régression des femmes dans l'arène de la représentation professionnelle ordinale, au demeurant, on observe que partout où la parité est une obligation, la place des femmes avancent et que quand ce n'est pas le cas, hé bien c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent. Pour ce qui est enfin de votre développement concernant l'ouverture de la possibilité de reconnaître un accès partiel un professionnel de santé communautaire problématique sur laquelle la ministre était intervenu et sur laquelle je suis intervenu dans mon intervention liminaire, hé bien, nous y reviendrons à l'occasion de la présentation du projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance l'ordonnance concernés, je vous remercie. Merci la discussion générale est Close, nous passons donc à la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, nous avons été saisis d'un amendement à la l'article unique sur ce texte pour le présenter, Monsieur Oui au nom de la mise en cohérence des textes 7 heures un ensemble de mettre un terme à un imbroglio juridique qui alimentait depuis plusieurs mois, les praticiens hospitaliers, suite à l'interdiction par la loi de modernisation de la santé des dépassements d'honoraires dans le cadre du service public hospitalier les praticiens hospitaliers du secteur privé ont critiqué l'autorisation maintenue pour les praticiens du secteur public de pratiquer une activité libérale à l'hôpital, l'ordonnance explicite donc l'articulation entre le principe de l'interdiction des dépassements d'honoraires au sein du service public hospitalier et le maintien d'une dérogation possible dans le cas de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein, alors que près d'un quart des Françaises et des Français renoncent ou reportent leurs soins dans l'année, principalement en raison des dépassements d'honoraires, la pratique de ces dépassements par des médecins, le pital doit être, selon nous, interdite et quelle que soit leur statut actuellement moins de 5 pour 100 100 des médecins exerçant dans les établissements hospitaliers publics pratiquent des dépassements d'honoraires, cette interdiction aurait donc un effet limité sur l'ensemble des praticiens, serait une mesure de justice sociale pour les patients les plus précaires et de lisibilité pour les patients qui ont du mal à distinguer, en effet, selon que le médecin exerce son activité en libéral au public afin de garantir une rémunération des médecins hospitaliers, l'ensemble des personnels de l'hôpital public, il est par contre nécessaire de mener une politique audacieuse de revalorisation de leur rémunération ainsi que du point d'indice. Merci, est ce qu'il y a de l'avis de la commission. chers collègues, l'ordonnance de mise en cohérence des textes au regard de la loi santé se contente d'expliciter le maintien possible d'une dérogation à l'interdiction des dépassements d'honoraires au sein du service public hospitalier dans le cadre d'une activité libérale, cette possibilité de paraît pas contradictoire avec le cadre établi par la loi santé dès lors qu'elle intervient dans des conditions précises, notamment, comme le prévoit l'article L 61 54 tiré 2 en garantissant l'information des patients et la neutralité de leur orientation, elle interroge toutefois, comme l'a souligné Macaulay Catherine Deroche sur la différence de traitement entre les établissements publics et privés à ce sujet, dans la mesure où les modalités d'application de ces dispositions sont renvoyés au pouvoir réglementaire, je demanderai l'avis du gouvernement sur la manière dont il entend mettre en 9 cette possibilité de dépassement d'honoraires. A l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Madame le rapporteur cette ordonnance ne procède à aucune modification substantielle de la loi, elles ont au contraire on apporter clarification, elle ne fait que suivre l'intention qui a été exprimée par le législateur, en effet, vous savez, la loi de modernisation de notre système de santé a réintroduit dans notre législation, la notion de service public hospitalier et ce afin donner davantage de lisibilité aux patientes et aux patients dans l'offre hospitalière, le service public hospitalier a ainsi été ouvert à l'ensemble des établissements de santé, indépendamment de leur statut, il repose non plus sur une liste de mission mais sur des obligations de service public qui s'impose aux établissements de santé, faisant le choix du SPA parmi ses obligations figurent notamment l'accessibilité financière et donc l'obligation de proposer à chaque patient de chaque patient, une prise en charge, sans dépassement d'honoraires, cette obligation n'est en aucune manière, remise en cause par cette ordonnance. cette obligation pardon n'est toutefois pas incompatible avec la possibilité pour les praticiens hospitaliers dans le respect, non sur des conditions posées par la loi de pratiquer les dépassements d'honoraires dans le cadre de leur activité privée afin de lever toute ambiguïté : l'ordonnance précise donc l'articulation entre les dispositions sur le service public hospitalier et celles relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers ces praticiens ne peuvent réaliser des dépassements d'honoraires que dans des conditions de gens précise et sous réserve que les patientes et patients puissent bénéficier d'une alternative sans dépassement d'honoraires l'activité libérale des praticiens hospitaliers est par ailleurs très encadré, le praticien doit au préalable, signer avec le directeur de l'établissement, un contrat d'activité libérale soumis à l'approbation du directeur général de la RS le directeur ou la directrice de l'établissement, la possibilité de s'appuyer sur les nécessités du service public pour refuser la signature d'un contrat d'activité libérale qui ferait obstacle à ce service, ainsi, contrairement à la situation qui est connu dans les établissements privés, ce régime n'est pas un droit absolu des praticiens cette possibilité de réaliser une faible partie de son activité à titre libéral contribue également à maintenir l'attractivité des centres hospitaliers publics et notamment des CHU pour les professionnels de santé et ainsi à garantir le maintien d'une offre d'excellence dans le service public hospitalier, enfin et surtout, cette activité reste très marginal dans l'activité dispensée au sein des établissements publics, elle ne concerne qu'un nombre faible de praticiens et de praticienne en 2014, seuls 10 pourcent des des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein étaient autorisés à exercer une activité libérale, parmi eux 2041 praticiens hospitaliers à temps plein, exerçait en secteur 2 soit environ 4 pourcent de de l'ensemble des médecins hospitaliers, l'avis du gouvernement et donc défavorable. Donc madame la porte, vous en retient l'avis du gouvernement. Donc 2 avis défavorables, il y a-t-il des explications de vote. Non, donc nous passons au vote qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient

Nous passons maintenant à la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 19 janvier 2017 relatives à la profession de physicien médical et l'ordonnance du 19 janvier 2010 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

c'est un moment de coordination ce président. Très bien, merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission sur l'article 2 du projet de loi ratifiant l'ordonnance

oeufs 4 amendements sur les articles additionnels. Le premier amendements. Après l'article 2 j'appelle raison qui va prendre la parole sur cet amendement, j'ai une longue liste de signataires. Je vais pas vous la cité. Monsieur Chevrollier peut-être monsieur Bouillet. est marqué que l'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestations de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, or la profession dans une Venise déplore une évaluation n'effectif de la maîtrise de la langue, c'est un amendement a vocation, a précisé que cette évaluation s'effectue au moment de l'examen de ces qualifications professionnelles et soit réalisée sur un outil qui pourrait s'apparenter au cadre européen commun de référence pour les langues appliquées aux professionnels de santé, voilà, il est l'objet de se présente amendements. Merci Monsieur le Président ne présente amendement propose une modification du code de santé publique, afin de garantir que la profession d'orthophonistes soit exercée en France par des professionnels, maîtrisant la langue française, il permettra de s'assurer de la maîtrise du français par l'orthophoniste demandeurs d'une reconnaissance de ces qualifications et de garantir ainsi la protection des patients et la qualité des soins dispensés. La Commission européenne, en effet, a elle-même reconnu la maîtrise de la langue comme compétence des orthophonistes et il serait donc nécessaire qu'elle apparaisse dans la transposition de la directive si la directive afférentes stipule que, je cite, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles, fin de citation, la Commission européenne confirme dans ces documents d'accompagnement à la mise en oeuvre de la directive code de conduite et guide de l'utilisateur, qu'il existe toutefois une exception Assad règle lorsque les connaissances de linguistique, font partie de la qualification ensuite l'exemple de l'orthophoniste ou du professeur enseignant la langue du pays d'accueil, il n'y a donc pas d'impossibilité de mise en oeuvre d'une telle disposition qui sécurisera davantage la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Merci, il y a des articles identiques qui suivent celui c'est monsieur Vatrin qui le défend. Oui, ben je vais pas tout reprend des arguments déjà été donnée mais je pense que le l'objectif de ces amendements, c'est de garantir aux patients souffrant de troupes du du langage en France des soins de qualité et que nous sommes d'accord tous pour dire que il est indispensable, dans ces conditions que les connaissances linguistiques soit intégrés et vérifier, or l'adoption de l'ordonnance en l'état, rendrait impossible de procéder à un contrôle a priori, alors on m'a dit que c'était pas vrai, ce matin en commission, j'ai donc regardé ce qui est marqué dans le code de la santé publique et c'est vrai que c'est pas clair, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il est marqué que l'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestations de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, donc ça règle pas notre problème si c'est a priori ou à posteriori mais si on regarde le texte de l'ordonnance elle-même, beaucoup moins ambigu et c'est très clair, c'est ce que c'est marqué ceci : le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionnée à l'activité exercée et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue, c'est donc un contrôle à postériori, contrairement à ce qu'on m'a dit ce matin donc, vouloir à tout prix transposer une directive européenne, sans s'occuper de ses conséquences, hé bien ce serait pour nous une erreur et même une faute car contraire à l'intérêt même des patients, mais vu l'intérêt la nécessité que les orthophonistes maîtrisent la langue française sur un sujet relatif au langage, c'est pourquoi nous vous demandons de voter cet amendement. Oui, dernière amendements identiques présentés par Madame Rossignol. Les 4 amendements qui ont été présentés lundi qui sont convergents, révèle qu'il y a pas d'minima un malentendu, au pire une incohérence juridique et une incertitude graves qui aboutit à ce que les professions d'orthophonistes sont inquiète sur la transposition de cette directive et j'ai entendu les arguments qui ont été développé d'abord par la ministre de la Santé au lors de la lecture à l'Assemblée nationale et puis ensuite ce matin en commission qui tendent qui tendrait à rassurer les orthophonistes, si tant est que vous lisant convainquez les uns et les autres, donc il me paraît indispensable pour lever justement ces malentendus incohérence ou incertitudes juridiques que nous ayons une explication extrêmement sécurisé sur cette affaire de connaissances Agusti qu'exiger a priori ou à posteriori pour l'exercice d'une profession comme celle d'orthophonistes où chacun comprend bien que la nature même de l'exercice de ce métier exige des connaissances parfaite de la langue, des enfants qui sont accompagnés, merci. Alors l'avis de la commission d'abord sur l'amendement de monsieur Perrin raison etc à rectifier lisse. Merci Monsieur le Président, tout d'abord quelques mots avant de donner la vie de de la commission, cette question fait effectivement partie de celles qui m'a largement occupé pendant les auditions, puisque j'ai en effet, été interpellé par les constatations concordantes de plusieurs professions de santé quant à la réalité de l'évaluation des compétences linguistiques des professionnels de santé européens souhaitant exercer en France, il semble en effet que cette évaluation soit faite de manière très différent d'une profession à l'autre et au sein même d'une profession de manière très différent d'une commission départementale ordinale à une autre, la Cour des comptes a d'ailleurs souligné cet inquiétant phénomène à propos de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, en soulignant que les commissions des départements les bien moins d'Otan professionnels médicaux pouvait se montrer plus souple, la question est pourtant d'une importance cruciale pour la qualité des soins dispensés aux patients, il me semble cependant que les amendements déposés ne permettront pas de répondre à cette préoccupation, je comprend à la lecture et notre collègue Vatrin l'a très bien exprimé l'inquiétude qui porte sur le fait que le contrôle de la maîtrise de la langue puisse intervenir à posteriori l'autorisation d'exercice accorder un professionnel non français, il me ce qui me semble, cependant, et vous avez cité le texte même de or de l'article que la rédaction proposée par la tactique, le 3 du projet de loi prévoit bien que le contrôle des compétences linguistiques interviennent effectivement une fois la qualification professionnelle reconnue, c'est-à-dire une vérification du diplôme, mais au moment de la délivrance de l'autorisation d'exercice, on fait le distinguo entre le la la vérification vérification de la qualification professionnelle et l'autorisation qu'il est bien distinctes le madame la ministre pourra cependant nous éclairer utilement sur son point sur ce point, en confirmant ou non cette interprétation, la question des qualifications linguistique n'est toutefois ne toutefois elle ne devrait pas être réglé par pardon, dans le cas de la loi qui prévoit des le principe d'une évaluation linguistique mais au stade de son application, le principal problème est en fait celui de l'harmonisation de ce contrôle, pour cela, les professionnels devant de santé devrait à mon avis, disposer d'un outil d'évaluation de référence qui aujourd'hui fait défaut, il pourrait d'ailleurs être adapté à chaque profession autour d'un trou commun il faudrait, en somme, que l'on dispose d'un test sur le modèle du taux unique avec un volet portant aussi sur la langue médical il appartient donc au gouvernement de mettre en place telle août donc, c'est une demande de retrait sinon un avis défavorable. C'est sur l'ensemble des amendements, les trois identique, madame la ministre. Merci Monsieur le Président, effectivement, la maîtrise de la langue française, fait déjà partie des qualifications professionnelles et elle nécessaire à l'exercice du métier d'orthophonistes, à ce titre, les commissions d'autorisation d'exercice opère d'ores et déjà ce contrôle en faisant procéder à une audition des candidates et des candidats si et quand elle estime nécessaire, le gouvernement et donc pas favorable à l'amendement proposé puisqu'il est déjà satisfait en réalité. Merci

Oui, simplement vous dire que je vote à l'amendement regardez explication donnée par un rapporteur et les précisions apportées pendant le ministre. Donc, il reste au vote 3 identiques qui ne sont pas. Retiré malgré la demande donc Madame le rapporteur. Nous passons au vote qui est pour ces amendements identiques.

Qui est contre. Qui s'abstient l'ensemble du projet de loi est adopté, je mets au voient l'ensemble du projet de loi non c'est bon, c'est : on a pris et là, dernier la discussion du dernier projet de loi ratifiant l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Allemande ment numéro 4. Je suis maire, Madame Imbert, pardon. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président. C'est un amendement rédactionnel excusez-moi midi l'avis du gouvernement sur le rédactionnel. avis favorable. Très bien, qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il était adopté, je mets au voix l'ensemble de l'article 2 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, article 3. Plusieurs amendements non un amendement de du gouvernement mais ministre. Merci Monsieur le Président, comme les médecins comme les chevaux jeunes chirurgiens dentistes souhaite assurer une représentation des praticiens exerçant en Corse au sein de la chambre disciplinaire interrégional de 1ère instance de Provence Alpes Côte d'Azur, Corse, en leur réservant un siège sur les 4 de cette instance, quel est l'objet de l'amendement qui est soumis à votre approbation. Merci Monsieur le président, madame la ministre, les 3 amendements, donc qui vont nous être présentées, dont celui que vous venez de présenter à l'instant été déposés tardivement hier, j'en ai eu connaissance dans sa rédaction ce matin seulement, donc, la commission n'a pas eu les moyens des expertises et néanmoins la clé de répartition des sièges proposés au sein de cette instance inter-régional Provence Alpes Côte d'Azur, Corse, vise à garantir une représentation équilibrée des professionnels issus des 2 régions concernées, cela semble être une précision raisonnable, même si on peut se demander pourquoi seuls 7 chambres interrégionales fait ainsi l'objet d'une telle clé de répartition de ces sièges c'est la spécificité, l'exception Corse, la Commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat en en rajoutant que nous avons tout de même pris la tâche du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas d'opposition à votre amendement. Y a-t-il des explications de vote. Je n'en vois pas hé bien donc sagesse de la Commission sur l'amendement du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Je mets au voient maintenant l'ensemble de l'article 3 il y a-t-il une explication de vote. Il n'y en a pas, qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté l'article 3 bis, pas de 2 explications vote non et je mets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté l'article 3 bis B. Même vote, vote article 3 bis ce c'est il y a je suis saisi. Un amendement de Madame le rapporteur madame Habert. C'est un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président. Merci. Le gouvernement son avis. Avis favorable du gouvernement surprise. Pas d'explication de vote la dessus donc nous passons au vote qui est pour. Qui et contre qui s'abstient, il est adopté, je mets au voix l'ensemble de l'article 3 bis, c'est qui est pour.

je suis saisi. Un amendement du gouvernement le moment numéro 3 madame la Ministre. L'ordonnance du 16 février 2017 a modifié, dans son article 10 la composition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le CNE à l'article L. 42 31 4 du code de la santé publique, les 2 représentants du ministère de la santé sont désormais désignés par le directeur général de l'offre de soin et le directeur général de la santé et assiste à toutes les délibérations avec voix consultative et l'article 19 de la même ordonnance a fixé l'entrée en vigueur de la nouvelle composition du CNO, à compter du prochain renouvellement du Conseil de l'Ordre suivant sa publication, ce qui est tardif, il y a donc opportunité à permettre une présence effective et immédiate de l'administration au regard des attentes formulées par l'Ordre des pharmaciens lui-même demandeur d'échange de consultation et d'information, il vous est donc proposé d'établir une date d'entrée en vigueur immédiate pour la disposition regardant spécifiquement les représentants de l'administration au sein du CNO, à compter de la publication du présent projet de loi de ratification, l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professionnels de santé, telle est l'objet de l'amendement soumis à votre approbation. Avis de la commission Madame le rapporteur. Merci monsieur le président, les dispositions fixant la composition du Conseil national de l'or des pharmaciens ont été modifiés successivement par la loi santé de 2016 puis l'ordonnance du 16 février 2017 pour rétablir rétablir la présence de représentants du ministère de la santé, avec voix consultative à l'exclusion de disciplinaire les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance de février 2017 conduire à ce que cette nouvelle composition entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de ce conseil qui doit intervenir en juin 2018 anticiper sa mise en 9 paraît là aussi raisonnable, la Commission s'en remet à la ce geste du Sénat en vous précisant, mes chers collègues, que l'Ordre des pharmaciens est au courant et n'a pas émis d'observation et que nous avons ce même dispositif à l'ordre avec l'Ordre des médecins. Donc, vote sur cet amendement du gouvernement a classé sagesse de la commission qui est il y a pas d'explication de vote. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, nous passons au vote de l'article

qui est pour. Contre qui s'abstient, il était adopté, je mets au voix l'ensemble de ce projet de loi ratifiant l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des hors des professions. Santé il n'y a pas d'explication de vote non qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, merci d'être adopté, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 17 Pour la la déclaration du gouvernement, suivie d'un débat sur l'avenir de l'Union européenne en application de l'article 50, tirée de la Constitution, la science est suspendu.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement, suivie d'un débat sur l'avenir de l'Union européenne, ceci en application de l'article 50 de notre constitution. En les accueillant avec plaisir, madame et monsieur le ministre, et pour ce 1er débat de ce nouveau Triana les président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées de la Commission pour l'Union européenne à qui je souhaite le meilleur dans leurs travaux, je vais maintenant donner la parole à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,

Merci monsieur le président, Monsieur le Président, Madame la ministre. Messieurs les présidents des commissions des Affaires étrangères des affaires européennes, la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs. L'Europe et le cadre primordial et naturel dans lequel nos valeurs et nos intérêts doivent être portés à l'heure de la mondialisation. Elle est le coeur d'un projet majeur pour la France. Le président de la République a fait de l'ambition européenne renouveler une priorité de son mandat pour la France, c'est ce qu'il a exprimé avec force d'abord à Athènes puis à la Sorbonne le 26 septembre dernier. En affirmant les 2 convictions qui ont guidé son action et celle du gouvernement depuis le 1er jour. La 1ère c'est que dans un monde en en proie aux crises et à des bouleversements sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Seule l'Europe nous permettra d'exercer pleinement notre souveraineté de conserver la maîtrise de notre destin. La seconde, c'est que le projet européen ne peut réussir si nous ne comprenons par le fossé qui n'a eu de cesse, depuis quelques années de se creuser entre les peuples et les institutions européennes, au risque de voir le populisme et un nationalisme dévoyé submergé notre démocratie comme celle de nos partenaires. Oui, l'Europe est le déterminant majeur d'une politique globale. pour que la France fasse entendre sa voix, il nous faut un cap clair, le président l'a fixé. Et vous avez entendu ses nombreuses propositions pour l'Europe. signez souligner devant vous, qu'elle s'articule autour de 2 horizons de temps : d'abord l'échéance de 2019 vous seront organisés les prochaines élections européennes, il faut nous y préparer, cela nous donne le temps de convaincre nos partenaires. 2019 donc 2024 ensuite, qui sera l'horizon de la nouvelle Commission résultant de ces élections et nous devons avoir pour objectif de lui proposer un mandat ambitieux porté par la volonté de refonder l'Europe. L'ensemble du gouvernement est mobilisé derrière le président de la République au service de ses objectifs. Et pour préparer au mieux ce rendez-vous. Il nous faut aussi une conscience lucide de la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Et en la matière, et alors que la défiance est installé dans une partie des peuples européens, rien ne serait pire que le déni de réalité, l'Europe est aujourd'hui perçue comme trop lointaine comme trop technocratique, incapable de rendre intelligible cette décision comme ses instruments de légitimité démocratique, elle suscite une forme d'indifférence résignée dont on a encore témoigné le faible taux de participation aux dernières élections européennes, et pour autant, nos concitoyens n'ignore pas l'Europe, en vérité, elle est revenue au centre de l'attention, mais trop souvent d'une manière négative. Avec des crises qui ont frappé le continent ces 10 dernières années, elle a été tantôt pointé du doigt en cas d'échec tantôt laissé dans l'ombre lorsqu'elle apporter des solutions, je ne crois pas que nous ayons assez dit ce que l'Union européenne rendait possible et ce qu'elle apporter concrètement à nos concitoyens, en outre, depuis 15 ans des forces centrifuges traverse le continent, elles ont atteint leur paroxysme avec la décision du Royaume-Uni, de quitter l'Union européenne. Cela il y a un peu plus d'un an. C'est la décision souveraine du peuple britannique et nous la respectons, même si elle représente une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Depuis le 19 juin la négociation est enclenchée, sous la conduite de Michel Barnier, il a reçu un mandat clair des 27 États membres de la Commission européenne sur la base des orientations arrêtées à l'unanimité par le Conseil européen en mai juin dernier. Je vous en rappelle les principes. Qui fonde la position des 27. Garantie réciproque pour les citoyens, directement concernés par le Brexit respect par le Royaume-Uni de ses obligations administratives, financières et juridiques souscrite en qualité d'États-membres prise en compte de la spécificité de la frontière irlandaise et y ajoute évidemment sur le marché intérieur, le rappel du caractère indivisible des 4 libertés de circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes. Je tiens aussi à préciser, mais vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, aucune négociation ni sur les conditions du retrait, ni sur les contours de l'accord futur ne saurait être mené à titre bilatéral. Il importe de le rappeler. Dans cette crise, l'Union européenne, fait la preuve de son unité et sa cohésion. Il ne s'agit pas pour autant d'adopter une n'approche punitive à l'égard du Royaume-Uni, le Renault munir restera après son retrait, un partenaire et un allié essentiel de la France, tout particulièrement dans le domaine de la défense, je tiens à le rappeler une nouvelle fois en vertu. Des accords de Lancaster House qui sont toujours présents et est garantie dans le cas de notre relation bilatérale, mais nous ne devons avoir par ailleurs aucune naïveté dans la négociation en cours. Chacun défend ses intérêts. Notre intérêt collectif, c'est de mettre fin dès que possible à l'incertitude que fait planer le Brexit et le faire en 2 temps d'abord en négociant les conditions du retrait et seulement ensuite en instaurant le cadre juridique de nos futures relations. Pour l'heure, après les premières sessions de négociations, force est de constater que le compte n'y est pas, s'agissant des différents principes que que j'ai rappelé et qui conditionnent pour nous un retrait acceptable du Royaume-Uni, le discours de Theresa May à Florence, il y a quelques jours à donner des signes d'ouverture, la 4ème session a permis quelques progrès mais il reste insuffisant, nous sommes dans la 5ème session en ce moment, compte prochain conseil européen qui se tiendra en quelques jours, ne pourra sans doute pas décidé d'ouvrir les discussions de la 2ème phase avec le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs les sénateurs hier le vote britannique. Ces derniers temps la défiance d'un nombre important de nos concitoyens. Aujourd'hui, la crise qui secoue la Catalogne en ce moment même. Tout cela nous commande d'agir. Nous ne pouvons plus nous permet de continuer à faire l'Europe, comme par le passé. Il faut revoir en profondeur nos priorités politiques, nos pratiques institutionnelles et les moyens qui sont dédiés à chaque objectif un sursaut. Une véritable fondation pour reprendre l'expression du président de la République sont indispensables. Je veux dire aussi. Ceux qui dénoncent aujourd'hui la construction européenne. Qu'ils entretiennent nos concitoyens dans une représentation chimérique de la souveraineté, la souveraineté de repli qui propose à nos concitoyens est à l'heure, elle ne peut mener la France qu'à l'isolement et à une Exposition plus grande encore notre pays aux désordres du monde. C'est une communauté destin qui nous uni aux peuples d'Europe. Dire cela, ce n'est pas faire l'aveu d'une fatalité, c'est affirmer à la fois une histoire partagée et une vision stratégique et volontariste de la place de la France dans le monde. Je suis en charge aujourd'hui de la conduite de la diplomatie de notre pays et je peux vous le dire, jamais depuis la fin de la guerre froide. Les divergences mais attention le niveau de conflictualité n'ont été aussi élevées. Dans un monde pourtant de plus en plus interdépendant, la compétition est à son paroxysme. La coopération entre nations, de moins en moins évidente. La multilatérale est en voie d'affaiblissement, les crises se sont multipliées dans le voisinage immédiat de l'Europe. Des stratégies de puissance affirme de façon de plus en plus agressive, la concurrence économique les tensions commerciales les inégalités que génère la mondialisation s'accroissent dans ce contexte, la seule réponse qui vaille est à la fois nationale et européenne, les 2 dimensions sont aujourd'hui inséparables et si la France veut garantir sa sécurité si elle veut défendre ses intérêts et affirmer ses valeurs, bref, si la France veut compter dans le concert des nations et continuer d'écrire par elle-même son histoire alors sa souveraineté passe par son effort propre et aussi par l'Europe mais une Europe réformé une Europe capable de s'affirmer elle-même comme une puissance souveraine. Pour faire entendre sa voix, l'Union doit donc intégrer une culture du rapport de force, je le redis une culture du rapport de force qui lui a trop souvent fait défaut. défaut. Il a dirigé les sénateurs cette Europe souveraine repose elle-même sur 3 conditions : d'abord l'unité de l'Europe, ensuite, la protection de ses citoyens et ses intérêts, enfin ce que j'appelle la capacité de projection de l'Union européenne, c'est-à-dire sa capacité à agir comme un acteur global à peser réellement sur les dossiers internationaux et à diffuser son modèle et ses valeurs. La première condition de l'Europe souveraine, c'est le renforcement de son unité. Mais ce travail d'unification est vouée à l'échec s'il ne prend pas réellement en compte les aspirations des peuples, dépositaire de la souveraineté européenne au peuple français. Les peuples d'Europe doivent être de véritables acteurs de cette refondation, si nous voulons qu'une authentique démocratie européenne existe. C'est la raison pour laquelle. La France propose l'organisation de convention démocratique dans tous les États membres qui souhaiteront participer à cette initiative, il s'agit de redonner la parole au au citoyen et de débattre sur le fond au plus près du terrain de débattre des priorités de l'Union pour les années à venir. Au 1er semestre 2018, chaque État membre qui le souhaite pourra déployer selon les modalités qui lui paraissent les plus adaptées, une série de débats et d'échanges dont les conclusions seront mis en commun pour préparer l'échéance de 2000 19 et refonder l'Europe en répondant mieux aux attentes des citoyens qui ont cette fois été consultés en amont. La ministre chargée des affaires européennes Nathalie Loiseau est mobilisée pour donner corps à ce projet de la façon la plus large possible avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs syndicaux de la société civile pour que ce soit une vraie mobilisation qui puisse mettre en oeuvre. Renforcer l'espace démocratique européen, le mettre en mouvement animé par un projet sachant dépasser les seules formations politiques nationales, c'est aussi le sens de la proposition du président de la République de créer une circonscription européenne. Les députés européens seraient élus sur la base de listes transnationales selon un principe simple : rassembler des candidats de même sensibilité politique mais de nationalité différentes. 7 circonscriptions transnationales, ce sera l'occasion toute particulière d'une réponse européenne au Brexit. L'unité de l'Europe, et bien sûr une réalité politique, c'est aussi une réalité économique, je vais y revenir, mais la base le socle sur lequel tous ces projets peuvent se construire. C'est le lien insensible le vivre-ensemble en un mot la conscience qu'ont nos concitoyens d'être des Européens. Fortifier cette conscience, tout particulièrement dans notre jeunesse par l'enseignement. Par les échanges universitaires et par les échanges d'apprentis, c'est garantir l'avenir de l'idée européenne c'est universel, qui se dit en plusieurs langues, cette civilisation que chacune de nos cultures nationales exprime d'une façon propre d'une façon singulière, un enjeu d'égalité notre jeunesse n'a jamais été aussi mobile aussi ouverte sur le monde et d'abord sur les pays européens, assurer une égalité d'accès à l'horizon européen, c'est aussi de cette manière que nous conjugueront l'unité de l'Europe et l'exigence démocratique. Les objectifs qu'afficher le président de la République sont ambitieux. Ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, doit pouvoir le faire sans en être en pêcher. Les coopérations seront ouvertes à tous, avec pour seul critère, le niveau d'ambition partagée. Le président de la République a d'ailleurs proposé. De réunir au sein d'un groupe de la refondation européenne tous les États-membres qui partagent cette vision afin de définir les mesures qui traduiront concrètement cette ambition à l'horizon 2020, je dois dire que l'accueil réservé à nos propositions par nos partenaires à la fois lors du sommet des chefs d'État ou de gouvernement à Tallinn. à la fois en déclinant les propositions portées par le président de la Commission, Jean-Claude Junker, à la fois par la volonté du président du Conseil donne Alta qui est aujourd'hui même à Paris, l'ensemble de de D accueil de ces différents acteurs, montre que la feuille de route qui va être initiée par le président Donald Teske pourra permettent d'aboutir dans cet exercice collectif de refondation. Pour avancer. L'Allemagne sera notre partenaire majeur. Vous le savez, la République fédérale est entré dans une période de négociations du contrat de coalition sous l'égide d'Angela Merkel. Je tiens d'ailleurs à souligner la qualité des relations qui sont ceux qui se sont nouées depuis plusieurs années entre les ministres allemand et les membres du gouvernement. Cette passe politique cette base relationnel est essentiel pour porter le projet européen, et cela est d'autant plus important. Que les élections allemandes, avec notamment le score très élevé, de l'extrême droite ont révélé que le scepticisme, voire le rejet de l'Europe était également un risque outre-Rhin. La meilleure réponse sera apportée par l'action conjointe d'Angela Merkel et des mêmes Macron pour permettre à l'Europe de progresser en puissance et de relever les grands défis qui nous font face, et de les relever dans la solidarité, nous avons été si souvent le moteur de l'Europe par le passé. Nous serons de nouveau demain le président de la République a souhaité l'élaboration d'un nouveau traité de l'Élysée, il pourrait être le creuset d'ici qui au projet européen. L'unité de l'Europe doit aussi se manifester face à la crise migratoire. Ce drame exige la solidarité des pays européens. Solidarité s'agissant de l'accueil du droit d'asile. Mais solidarité aussi dans l'aide à apporter aux pays de Transit. Pour éviter que. Ceux et celles qui font l'objet de tentation des passeurs ne risquent leur vie pour rejoindre l'Europe, c'est dans ce but que le président de la République a réuni à Paris le 28 août dernier ses homologues allemands, espagnols tchadien, nigérien ainsi que la haut de représentants de Federica Mogherini c'est aussi le sens des mesures concrètes. Que le président a exposé, dans son discours de la Sorbonne, je pense à la mise en place d'un véritable office européen de l'asile pour harmoniser les procédures. Je pense aussi à la création d'une police aux frontières européennes sur ce sujet comme sur d'autres. L'exigence de solidarité européenne repose sur un équilibre. Sur une réciprocité entre les droits et les obligations. La cohésion entre les États et la cohérence du projet européen comme sa légitimité passe par là. L'unité de l'Europe passe également par une convergence sociale et fiscale accrue. Jacques Delors a coutume de dire. Que le modèle économique européen doit se fonder sur 3 principes : la concurrence qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui réunit, force et la solidarité qui réunit, force est de reconnaître que l'Union européenne a davantage annoncé sur le 1er volet que sur les 2 autres, or il est fondamental de préserver un équilibre pour que les États-membres converger économiquement et socialement, et le fasse vers le haut, c'est ce que nous demandons, nos concitoyens, notamment au travail détaché. Je sais que ce sujet mobilise l'attention et le travail du Parlement. La directive actuelle n'est satisfaisante pour personne, ni pour les travailleurs français qui font face à une concurrence déloyale. Ni pour les travailleurs étrangers dans les conditions de vie et de travail sont souvent insuffisamment protectrice, ni pour leur pays d'origine, qui souffre d'une insuffisance de Madoff qualifié l'ensemble des ministres concernés par ce dossier et mobilisé avec une méthode claire parler à tous. écoutez nos partenaires. Notamment les pays d'Europe centrale et orientale afin de dégager des convergences avec le plus grand nombre d'entre eux Que la convergence sociale passe aussi par la définition d'un socle minimal des droits sociaux européens parvenir à cet objectif est indispensable, ça fait partie de la refondation et le 1er ministre participera à ce sujet à une rencontre à Göteborg, dans les jours qui viennent, pour nous permettent d'avancer. Cet objectif de convergence des niveaux développement c'est aussi le but du fonds de cohésion qui bénéficie aux États-membres les plus éloignés du niveau moyen de développement en Europe, il s'agit d'un outil puissant nécessaires pour minimiser les disparités entre les régions, un outil qui, en même temps, profite à la croissance collective. Et c'est le même objectif de minimiser ces disparités au sein de l'Union qui guide l'affectation des des fonds structurels, vous savez que la France bénéficie sur la période 2014, 2020 de 27 milliards d'euros au type de différents fonds et les élus que vous êtes savent l'importance de ce soutien européen à notre politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Sur le terrain économique, la condition de l'unité européenne, c'est bien sûr le marché unique. Avec un objectif aujourd'hui progresser sur l'union économique et monétaire en poursuivant l'établissement de l'Union des marchés de capitaux afin de stimuler la croissance, en favorisant l'investissement et l'innovation, de même, les discussions doivent se poursuivre sur l'achèvement de l'union bancaire avec la mise en place d'un système européen de garantie de dépôts. Plus généralement. Nous devons faire de l'Europe une véritable puissance économique et monétaire et c'est pour ça, de raisons. Donc le gouvernement porte une ambition forte pour la zone Euro. Nous souhaitons ainsi la renforcer pour qu'elle puisse tout d'abord mieux garantir ses membres contre les crises financières lorsque c'est nécessaire. La proposition du président de la République de créer un budget de la zone Euro constitue un objectif pragmatique au service, cette ambition. Le renforcement de la zone Euro nécessitera également d'inventer une gouvernance adaptée, avec un ministre comme un contrôle parlementaire au niveau européen, devant lequel il devra rendre compte et, plus encore qu'une gouvernance, il sera nécessaire de définir les grandes orientations économiques et politiques de la zone Euro. Pour lui permettent de s'affirmer comme une puissance économique mondiale capable de défendre les intérêts des États-membres, c'est exigence de protection que l'on retrouve là, c'est finalement le 2ème élément qui défini aujourd'hui, notre ambition d'une Europe souveraine. Le souci de protection. Il est inhérent au projet Euro européens y compris danser politiques les plus anciennes et les plus emblématiques, en effet, quelle était la préoccupation des Européens en instituant la PAC, c'était la protection du revenu des agriculteurs, la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. à ces objectifs historiques se sont ajoutées la protection de l'environnement et le développement rural et nous devons, dans le cas d'une part, de rénover nous assurer que ces objectifs essentiels seront encore mieux atteint pour que notre agriculture, assure un niveau de vie décent aux producteurs pour que les consommateurs puissent accéder à AT produits agricoles de qualité à un juste prix par ailleurs. Pour parler de la protection, la création du Fonds européen d'aide aux plus démunis a permis à la France de recevoir sur la période 2014, 2020, 500 millions d'euros pour la fourniture d'aide alimentaire aux plus démunis, cela représente pour les associations qui agissent dans ce domaine un quart de leur fonctionnement et de leurs frais d'intervention. Dans une mondialisation aujourd'hui perturbée par la concurrence entre grands blocs économiques. Et les tentations isolationnistes. Une Europe qui protège. C'est aussi une Europe qui cesse d'être naïve dans le domaine commercial. Nous progressons dans ce domaine. Je veux saluer la décision du Conseil européen de se doter d'une nouvelle méthode de calcul des distorsions de marché résultant d'intervention de l'État dans les pays tiers. S'agissant de la lutte contre la concurrence commerciale déloyale, nous veillerons à ce que la Commission fasse pleine usage de ce nouvel instrument anti-dumping en vue de défendre l'industrie européenne. Et, plus largement, nous devons refonder la politique commerciale européenne. Les négociations commerciales ne peuvent plus être menée porte fermée. Elles doivent être transparentes. Et ne peuvent plus concernait seulement les tarifs et les tonnages. Elles doivent pleinement garantir le respect des normes sanitaires et environnementales et contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et je le dis devant votre assemblée. Les accords de demain doivent être plus complet. Que ne l'est le CETA. Comprenons-nous bien, cet accord est un bon accord. Pour les ouvertures de marchés qui l'autorisait parce qu'il prévoit un véritable mécanisme juridictionnel de règlement des différends sur les investissements mais. Il doit être complété par un instrument complémentaire dans le Maine climatiques en particulier, c'est la voie choisie par le gouvernement est en outre le Parlement sera informé à chaque étape préparatoire de la ratification du CETA je parle là du CETA, mais une fois engagé d'autres accords ces accords devront être menées dans la plus grande transparence, c'est la raison pour laquelle le président de la République a aussi proposé que soit rapidement mis en place un procureur commercial au niveau européen, chargé d'assurer la protection de nos intérêts face aux pratiques commerciales litigieuses qui sont à l'oeuvre en permanence dans les échanges internationaux. Et parce qu'une puissance doit définir ses intérêts stratégiques. La souveraineté de l'Europe passe également par la sauvegarde de ses intérêts économiques majeurs le président de la Commission Jean-Claude une guerre, a présenté à la suite de son discours sur l'état de l'Union, une proposition visant à établir un cadre pour la surveillance des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques au sein de l'Union. Aujourd'hui, certains États membres comme la France sont dotés de dispositifs performants, d'autres mécanismes nationaux le sont moins. Certains États n'en ont aucun une coordination européenne est indispensable dans le cadre du marché unique. L'Europe de la protection. Sentant également sur le terrain de la défense et la sécurité. Je vais rappeler les crises internationales affecte nos intérêts dans les zones toujours plus proche de l'Europe, la Syrie, la Libye Sahel l'Ukraine. Sont à proximité ou à nos portes. Avec des effets Directs sur l'ensemble des pays européens génère la menace terroriste, elles font craquer les frontières de Schengen où vaciller l'architecture de sécurité européenne. Cette situation exige que nous soyons collectivement capables de définir ensemble nos intérêts fondamentaux de sécurité. La France en raison de ses capacités en raison de son engagement doit être à l'initiative d'abord. Dans la manière dont nous définissons nos propres intérêts nationaux en relation avec la souveraineté de l'espace européen avec l'Allemagne, nous avons aussi un partenaire qui est de plus en plus consciente des menaces diverses qui pèsent sur l'Europe. à l'Est comme sur son flanc sud et on l'a vu d'ailleurs récemment en Afrique, nous pouvons donc aussi sur ce terrain avancée avec la la définition d'une doctrine stratégique commune européenne. C'est la condition sine quoi, non de la mise en 9 de l'autonomie stratégique européenne, c'est en effet à partir d'une conception partagée de ces intérêts communs. Nous pourrons définir les capacités, le budget et la culture de sécurité commune qui donneront corps à cette dimension fondamentale de la souveraineté européenne s'agissant de l'Europe de la défense, vous le savez, 2 avancées majeures ont été récemment enregistré d'abord le projet de coopération structurée permanente qu'on appelle généralement CSP, sur la base d'une contribution. Proposée par la France il y a un an, proposé par la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais soutenu aussi par la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Finlande, la République tchèque. Sur la base de cette contribution une liste précise de critères à remplir pour participer à la CSPI a été établie, a été approuvée, assortie d'un mécanisme de vérification permettant de garantir que les critères ambitieux qui ont été fixées par la la coopération structurée permanente soit respecté par les États-membres désireux d'y participer. Les États de la CSP s'engage à fournir un effort particulier en terme de développement. S'engage à mettre à disposition des unités de combat pour des missions communes s'engagent à renforcer leurs capacités de défense, il appartient désormais à ce moment aux États-membres qui le souhaitent de notifier leur volonté d'y participer et de démontrer qu'il respecte les critères que nous avons fixé collectivement et ce. Avant la fin de l'année, le 2ème aspect des avancées dans le domaine de la défense connaissez aussi, c'est la proposition par la Commission de créer un programme européen pour le développement de l'industrie de défense, qui doit financer les investissements nationaux dans la recherche dans le développement de prototypes dans l'acquisition d'équipements et technologies c'est une avancée considérable. Les négociations sur ce programme sont en cours, c'est ce qu'on appelle le Fonds européen de défense. s'il est souhaitable que ces négociations aboutissent avant la fin du 1er semestre 2018 et l'enjeu sera alors de doter ce fonds de financement suffisant, mais les perspectives devront devront être négocier dans le cadre financier pluriannuel ils pourront atteindre 500 millions d'euros par an, c'est le chiffre qui sont avancés et on voit bien qu'il s'agit là d'un saut qualitatif tout-à-fait significatif. Mesdames et messieurs les les sénateurs. Le président a exposé par ailleurs les principales clés d'une Europe souveraine à construire. Outre la sécurité, il a cité la maîtrise des flux migratoires, la stabilisation de son voisinage la confirmation d'une transition écologique efficace et équitable l'affirmation en tant que puissance d'innovation en particulier numérique et la puissance économique et monétaire sur toutes ces politiques structurantes. Le président de la République a fait des propositions opérationnelles, vous les avez entendu il y a proposé à la fois sur chaque point, une vision et des projets concrets dans chacun de ces domaines, l'objectif est de construire une Europe capable d'agir comme puissance globale, c'est la 3ème dimension de l'Europe souveraine que j'évoquais en commençant sa capacité de projection. Je pense notamment à l'action que nous devons mener à l'échelle européenne, s'agissant de la régulation de la mondialisation et des inégalités qu'elle génère. Le sentiment d'être laissés pour compte et partagée par une part croissante des citoyens européens, l'espérance du progrès social qui a animé une société mal en point cette perception qui est aussi entre le désenchantement et la colère affecte profondément notre vie démocratique et elle met au défi les responsables politiques de proposer un chemin qui fait le pari de l'optimisme du progrès de l'ouverture, plutôt que de l'isolement, du repli et du déclin. Ce que nous citoyens réclament ce n'est pas un projet irréaliste une sortie de la mondialisation, c'est une mondialisation organisée selon des règles justes et équitables. L'Europe est un acteur économique de 1er plan de même niveau que la Chine ou les États-Unis et la donc des arguments à faire valoir dans les instances internationales pour agir en faveur de cette régulation que nos clubs réclament, sous réserve qu'elle soit unie et sous réserve qu'elles soient déterminées, de même, elle doit agir pour le développement économique et humain, en particulier en Afrique et de ce point de vue, l'Alliance pour le Sahel lancée cet été avec l'Allemagne et l'Union européenne a valeur d'exemple cet effort sera poursuivi. Avec la proposition du président Macron de reprendre les travaux sur la mise en oeuvre d'une taxe sur les transactions financières dont le produit serait intégralement affectée au développement. C'est aussi le cas s'agissant de la lutte contre le réchauffement climatique. Et la lutte pour l'environnement dans ce domaine, l'Europe doit être exemplaire. Elle doit être exemplaire pour convaincre à l'échelle mondiale, c'est le sens de la proposition de travailler à un juste prix du carbone et à l'instauration d'une taxe aux frontières extérieures de l'Union pour compenser le différentiel d'ambitions environnementales pour les entreprises les plus exposés à la concurrence internationale, on peut observer par ailleurs que la méthode d'action pour assurer un consensus des États autour de l'accord de Paris, en dépit de la décision américain. De retraite, trouvant là encore que la voix de la France porte lorsqu'elle est bien coordonner avec nos partenaires européens. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'Europe, ce sont des valeurs. Celle de la démocratie. L'Europe, ce sont des droits et des libertés publiques, l'Europe, ce sont les valeurs de paix et de coopération, et dans un monde en proie aux incertitudes. La volonté d'ouverture à laquelle le président de la République invite l'Europe répond à une exigence de responsabilité. L'unité, la protection, ce sont les conditions pour que l'Europe puisse se projeter et contribuer efficacement à la stabilité de l'ordre international pour que les normes qu'elle incarne soit un modèle crédible à l'échelle du monde. Pour la régénération qui naît aujourd'hui à la conscience politique. L'idée européenne passe pour une évidence. Nous pouvons nous en réjouir, bien sûr, tant ce sentiment illustrent les 70 ans de silence des armes que le projet européen rendu possible entre nos états. Grâce à une construction bâtie sur l'idée de réconciliation et qui reste la meilleure garantie de paix comme le rappelait sans cesse Simone Veil. Mais si nous voulons bâtir l'avenir de l'Europe, nous devons aussi nous rappeler que les créations humaines n'apparence n'plus assurée peuvent être balayés par les fracas de l'histoire, voir la folie des hommes. La valeur de la construction européenne. Cette création politique unique mesurons la non seulement en des termes de succès économique. Mais aussi en la ramenant à son origine, celle des drames du siècle passé et de la volonté qui permit l'était passé chacune des générations de notre pays peut rattacher la naissance de sa conscience européenne à un événement marquera un projet fédérateur. Je pense aux ruines de la guerre dans notre pays, s'est relevé aux premiers efforts de réconciliation avec l'Allemagne dans une Europe alors divisée par la guerre froide, je pense à la liesse lors de la chute du mur de Berlin, où l'émotion immense de voir Helmut Kohl et François Mitterrand, main dans la main devant l'ossuaire de Douaumont je pense. Au projet, la concrétisation de la monnaie unique Mesdames et messieurs les sénateurs, elle sera pour notre jeunesse, elle qui incarne l'avenir de l'idée européenne et qui devra en assumer demain la responsabilité, elle sera pour elle l'événement le projet à partir duquel elle fera sien l'idéal européen, c'est la question à laquelle nous devons répondre collectivement par notre détermination et notre action. L'horizon de notre souveraineté est européen, c'est en construisant avec l'ensemble des États membres de l'Union une une n'Europe s'ouvrait n'que nous assumerons nos responsabilités à l'égard du peuple français je vous remercie. Merci monsieur. Dans la suite du débat, la parole est à notre collègue André Gattolin pour la République en marche et il a 6 minutes. Minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, madame la ministre chargée des affaires européennes mais, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire mon immense satisfaction quant à la tenue ici de ce débat sur l'avenir de l'Union européenne des débats en séance publique sur l'Europe, nous en avons assez RAGU régulièrement, mais il ne rassemble en général il y a plus d'une vingtaine de sénateurs, bien loin de l'affluence d'aujourd'hui, ces débats ont habituellement lieu à la veille de chaque sommet européen en présence du secrétaire d'État aux affaires européennes, sur le fond nous égrenant à cette occasion un ordre du jour prévisionnel pléthorique, renvoyant à une multitude de points assez hétérogène qui ressemblent plus en fait à une liste à la Prévert qu'un véritable panorama de l'état de l'Union, c'est donc, je crois, une excellente chose que nous ayons donc enfin un débat générique sur l'avenir de l'Europe et je trouverais Monsieur le Ministre, particulièrement pertinent si vous l'acceptiez d'annualiser ce rendez-vous important pour l'Europe en militant de l'Europe, que je suis depuis plus de 35 ans je vous ne cache pas non plus la joie que me procure, monsieur le ministre, votre présence à ce débat, ainsi que le nouvel intitulé de votre ministère, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la tribu réalité de mon langage mais je trouve que ça quand même plus de gueule et surtout plus de sens que ministère des Affaires étrangères et du développement international n'est qu'une attitude qui n'est pas si ancien que ça et qui dénote une époque où on avait l'Europe discrète pour ne pas dire l'Europe honteuse dans ce pays, ce nouvel intitulé du Quai d'Orsay n'est pas qu'un symbole, mais il est le fruit, je crois, de la volonté d'un président français qui a, contrairement à ses plus récents prédécesseurs la matrice et la fille européenne viscéralement ancré en lui, grande audace d'Emmanuel Macron, ce fut d'avoir osé mettre l'horreur au coeur de sa campagne présidentielle et ce à un moment où notre pays comme notre continent était traversé par une succession de crises majeures, son audace original, ce fut donc d'avoir osé présenter l'Europe non plus comme une contrainte, mais comme un véritable atout pour notre pays et sa force politique aujourd'hui en tant que président en exercice, c'est de ne cesser de parler d'Europe, de parler à l'Europe et pour l'Europe, la persévérance européenne du président n'est pas discutable et son discours de la Sorbonne du 26 avril dernier ne serait être plus comme une fulgurance d'un jour qui remis serait la question européenne au rang des dossiers à nos ressortir qu'à la veille des prochaines j'ai séance européenne non ce discours important qu'il soit et il voulait s'inscrit dans une série d'interventions majeures d'Emmanuel Macron, avant et après son élection sur la centralité de l'enjeu européen pour notre pays et à ceux et à celles qui s'étonne de sa volonté pragmatique, exprimé à la Sorbonne, d'aller de l'avant, quitte à avancer, d'abord avec un groupe d'États volontaires pour déverrouiller le blocage institué par la règle de l'unanimité sur les défis aujourd'hui les plus capitaux que nous devons affronter, je les renvoie à la lecture de son discours du 18 avril 2016 à Bruz devant le collège de de l'Europe, qu'il était encore ministre et qu'il venait tout juste de lancer le mouvement en marche à celles et à ceux qui s'étonnent de voir l'importance primordiale qu'il accorde à la construction d'une défense d'une véritable politique de sécurité commune, je renvoie au grand meeting d'Emmanuel Macron du 19 avril dernier à Nantes à 4 jours du 1er tour de la présidentielle où je crois Monsieur le Ministre, que nous étions tous les 2 présents enfin à celles et à ceux qui s'étonnent de son propos à la Sorbonne, merci cher ami sur la souveraineté européenne et sur la reconquête de ne souveraineté nationale dans et par l'Europe en même temps que de son affirmation de l'urgence démocratique à mettre en place dès le 1er semestre 2018 des conventions démocratiques visant à définir avec tous les citoyens d'Europe, le cap à donner à l'Union pour les prochaines années, nous renvoyons au discours du président prononcée le 7 septembre dernier à Athènes à Athènes, où il a également affirmé sans souhait de voir instaurer des listes transnationales dès les prochaines européennes de 2019 l'idée en soi des bonnes nouvelles et le Parlement européen avait échoué à la poser à l'occasion des européennes de 2014 alors la vieille formation politique nationale même grimée en pseudo-partis européens ont la vie dure, en particulier en France où la question européenne semble être une chose pro-sérieuse pour être abandonnée à des élus qui pense Europe et qu'il agisse véritablement en européen mais le fait que ces propos de scission soit aujourd'hui portées par le président d'un des principaux États-membres de l'Union rend assez difficile sa mise à l'écart d'un simple revers de main, il n'y aura pas mes chers collègues d'Europe si nous ne sommes pas capables de faire émerger non pas une classe européenne mais une représentation politique de classe européenne dans l'ensemble des États-membres, un des plus grands succès de l'Union au cours des dernières décennies a été et demeure sans conteste le programme Erasmus, hé bien, mes chers collègues, il est grand temps d'instaurer un Erasmus de la rescousse représentation politique en Europe être député européen ne saurait se réduire à une commutation, Paris, Bruxelles ou Paris, Strasbourg, de même être parlementaire national avec toutes les prérogatives de contrôle et de transposition de directives européennes dont nous disposons, vous avez qu'à venir à la commission des affaires européennes, vous le sauriez chers amis supposerait une part significative d'entre nous accepte de détachés pour une durée d'au moins 3 mois au cours de leur mandat, soit dans un autre Parlement national soit au sein du Parlement européen de cette appréhension très concrète d'une autre culture politique de l'Union, je crois que notre représentation nationale gagneraient en agilité européenne et donc on influence réelle sur la manière dont l'Europe, notre Europe se construit en conclusion, ce n'est donc pas mes chers collègues, à un enlèvement d'horreur comme cela est écrit, mais à un élève au moment de la France par l'Europe et pour l'Europe, auquel le président Macron nous convie, nous aurions tort, je crois, de ne pas relever le défi qui nous est fait, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant notre collègue Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 7 septembre devant le Parthénon symbole éternel de la sagesse grecque sur la Pnyx Colin, de l'exercice de la démocratie athénienne 1er, gouvernement du peuple par le peuple, le président Macron à poser cette question : qu'avons-nous fait nous de la démocratie, 60 ans après le traité de Rome, le bilan est en effet mer partout en Europe, les droits de l'homme régresse, alors qu'ils étaient considérés par les traités, non seulement comme le fondement des institutions européennes, mais aussi comme le principe régulateur des relations avec nos avec nos voisins, au sein de l'Union des droits fondamentaux sont bafoués, qu'il s'agisse de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse des libertés académiques des droits des syndicats des minorités ou de ceux des femmes, alors qu'en juin dernier, notre communauté nationale s'est retrouvée unie pour célébrer l'oeuvre accomplie et le message délivré par Simone Veil, grande figure européenne qui fait notre fierté l'accès libre des femmes au droit à l'intervention volontaire de grossesse est menacé dans plusieurs des États-membres et de plus en plus entravées dans notre pays même, comment ne pas s'indigner en pensant à l'opprobre jeté à la face de celles et ceux qui ont choisi d'offrir le don d'amour à une personne du même sexe, que dire de la honte qui nous accable en pensant au triste sort que nous avons réservé à nos soeurs et nos frères en humanité, fuyant la terrible guerre qui ravage à nos portes, la Syrie, pays avec lequel nous partageons pourtant une frontière, la semaine dernière, l'Europe a offert au reste de l'humanité, le spectacle affligeant du sang versé pour empêcher les citoyennes et des citoyens de voter la Commission européenne justifie son lourd silence complice par son obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre, elle a été beaucoup moins neutre quand il s'il s'agit d'imposer au gouvernement grec de baisser les pensions de ces retraités les plus pauvres, la solvabilité de la dette passe avant la défense du droit de vote, pourquoi continuer d'ignorer dans le continent le plus riche de la planète, la misère croissante de celles et ceux qui sont privés de travail, qui n'ont plus de toit qui ne peuvent plus se soigner et qui viennent chaque jour grossir les files des soupes populaires comme aux heures les plus sombres de notre histoire européenne, allons-nous effacer encore longtemps de nos consciences humaines la pitoyable existence de celles et ceux qui travaillent le jour et dorment la nuit dans leur voiture en Allemagne dans ce pays que vous ériger en modèle pour une Europe que vous appelez de vos voeux des des salariés ont un salaire mensuel inférieur à 980 euros pis près de 5 millions d'actifs vivent avec moins de 450 euros par mois cette misère sociale, cette incapacité croissante des salariés à vivre dignement des fruits de leur dur labeur attise les braises de l'extrémisme et pousse les électeurs vers des partis anti-démocratiques raciste et xénophobe, pour la première fois depuis la guerre 94 députés Nazis vont siéger sous la coupole du Reichstag, entendez ce coup de tonnerre d'un orage à venir qui pourrait être bien plus terribles aujourd'hui vous nous proposez d'appliquer à la France ses vieilles recettes en instaurant un gouvernement économique de la zone Euro, totalement soumis aux critères de l'ordo, libéralisme allemand vous voulez priver notre Parlement de ses prérogatives budgétaires pour les confier au gouvernement des techniciens parce que vous jugez qu'en cette matière, il est toujours plus efficace de donner le pouvoir à des personnes qui ne le détiennent pas du Peuple. Quelle est la puissance des dogmes qui vous aveugle et vous empêche de reconnaître que la prix qualité sous le joug de laquelle vous assujettis c'est dépend toujours plus important de nos sociétés, nous conduisent à l'abîme, comment ne pas comprendre que les peuples refuseront maintenant d'être dépossédés de leur souveraineté au profit d'instances non élues, qu'il juge responsable de la dégradation de leurs conditions matérielles oui nous pensons avec vous qu'il faut refonder l'Europe, mais par pitié sur d'autres bases et avec d'autres principes que ceux qui aujourd'hui condamnent l'idée européenne dans son essence même offrait au peuple l'utopie mobilisatrice d'une république universelle, démocratique et sociale, un grand rassemblement des femmes et des hommes libérés de la peur du lendemain, rassurés sur leurs conditions d'existence et disponible pour travailler ensemble à l'avènement d'une nouvelle République, retrouver l'esprit qui anima jadis la démocratie athénienne pour laquelle l'exercice du métier de citoyens imposer l'apport de vivre bien ensemble je conclurai par ces fortes paroles de Victor Hugo, notre collègue qui siégeaient à la gauche de cet hémicycle à la place, aujourd'hui occupé par Madame Assassi en 1860 depuis son exil refusant la soumission à la dictature de celui qu'il appelait Napoléon le Petit, il déclarait : je le cite oh mes frères en humanité, c'est l'heure de la joie et de l'embrassement mettons de côté toute nuance exclusive à cette tout dissentiment politique petit en ce moment à 7 minutes sainte, nous nous sommes fixons uniquement nos yeux sur cette oeuvre sacrée sur ce bus solennel sur cette vaste Aurore les nations et confondons toutes nos armes dans ce cri formidable digne du genre humain, vive la liberté. Merci mon cher collègue. La parole est maintenant notre collègue Philippe bonne Carrère pour le groupe de l'Union centriste et pour 8 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le ministre, Madame la Ministre, chers collègues débattent de l'avenir de l'Union européenne c'est débattre de notre propre avenir de celui de tous les Français, c'est donner une vision et un espoir pour les générations à venir quantifier la conscience de nos concitoyens d'être européen, pour reprendre une formule que vous avez utilisé, monsieur le ministre, il y a quelques minutes, c'est aussi retrouver l'esprit qui a guidé les pères fondateurs de notre union lors de la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à proposer une refondation de l'Union européenne, force est de constater que depuis son élection, le président de la République ne s'est pas ménagé sur ce dossier et je souhaite saluer sa détermination, ainsi que le contenu des 2 discours ambitieux qu'il a prononcée début septembre à Athènes et il y a 2 semaines à la Sorbonne, le président de la République a posé les bases de son engagement et de son ambition pour l'Europe, pour retrouver le souffle originel de l'Europe, 2 piliers solides me paraissent important à mettre en exergue à une Europe plus démocratique devrait permette de renouer le lien avec les citoyens européens, deuxièmement, une Europe plus protectrice doit assurer un rôle concret aux institutions de l'Union dans un 1er temps il apparaît une volonté de recréer une Europe souveraine, unie et démocratique comme énoncé dans le discours de la Sorbonne, cette refondation démocratique ne pourra se faire qu'à nos souciant l'ensemble des citoyens à la réflexion et aux décisions à prendre, nous ne pouvons plus jouer entre guillemets avec l'opinion publique, comme cela était souvent le cas lors des décennies écoulées en particulier après différents référendums plus ou moins conclure, le président de la République a proposé que soient organisées des conventions démocratiques en 2018 dans l'ensemble des membres qui le souhaiteraient, afin d'écouter, de faire débat, que les Européens ont neutre la reconstruction doit partir du pape, c'est le meilleur moyen de donner l'envie d'Europe, c'est aussi une bonne manière d'intégrer des idées nouvelles, soutenus par les citoyens, je pense aussi que les parlements nationaux auront toute leur place dans ces conventions, il sera important que notre commission Monsieur Bizet, Monsieur le Président, contribue à ces débats et nous savons, monsieur le président, Gérard Larchet pouvoir bénéficier de votre soutien, nous avions produit l'année dernière un important rapport avec nos collègues des Affaires étrangères, intitulé pour relancer l'Europe, retrouver l'esprit d'Europe, il pourrait servir de base à une réflexion qui s'inscrit dans le cap, cadre des propositions du président de la République, redonner du sens à la démocratie européenne c'est aussi redonner une légitimité au Parlement européen, la proposition de listes transnationales aux prochaines élections européennes va dans le bon sens, elle améliore le sentiment d'appartenance à une communauté de citoyens européens la possibilité de partager un projet cela devrait peut-être également passer par un rééquilibrage des pouvoirs entre les différentes institutions communautaires avec un Parlement plus représentatif et plus démocratique, comme je l'évoquais il y a quelques secondes vous connaissez aussi l'importance de la question des moyens du montant du budget européen et la possibilité de disposer ou non dans le budget de la zone Euro, étant donné l'état de l'opinion publique et ce depuis de nombreuses est il y a urgence ces débats les 2 à venir seront je l'espère, celle de la reconstruction démocratique notre pays en sera acteur, il est revenu dans le débat, il a retrouvé ce que j'appellerais une volonté d'Europe, une exigence de responsabilité pour reprendre là aussi une un propos de l'intervention de Monsieur le Ministre, dans un second temps, et au-delà de la refondation démocratique de l'Union, il nous faut lui redonner du sens à la mesure de sa dimension, il y a la mesure des attentes des citoyens et j'entends à cet égard que nous, tout n'est pas non plus petit économies sur ces sujets pour cela l'axe principal sur lequel je souhaite m'a tardé et celui d'une Europe qui protège la protection peut couvrir défendent naturellement divers, une Europe qui protège, chers collègues, c'est une Europe qui tend vers une convergence des droits sociaux, des droits des salariés et de la fiscalité à cet égard l'initiative lancée par la France sur la révision de la directive dite des travailleurs détachés assez différente de ce que j'ai entendu il y a quelques secondes, elle est aussi bien sûr un marqueur fort aujourd'hui, la situation n'est pas convenable, tant pour les salariés que pour les entreprises, tant sont déséquilibrés, les conditions de travail et protection sociale dans ce domaine, nous devons également nous lancer ce qui est aussi une réponse à ce que nous avons pu entendre dans l'intervention précédente dans une refonte des bases de la fiscalité des entreprises, la convergence fiscale doit être recherchée pour limiter dans ping entre les différents États-membres, elle doit aussi nous permettent de nous protéger des stratégies qui ont à la fois en caractère d'optimisation fiscale mais qui ont aussi un caractère anticoncurrentiel de certaines multinationales vous avez reconnu la bien entendu la problématique propre à ce que nous appelons aujourd'hui les une Europe qui protège, c'est une Europe favorable au développement économique, à la recherche, à l'innovation technologique mais c'est aussi une Europe suffisamment unie et puissante pour adopter des règles justes vis-à-vis de ce type d'entreprises qui ne peuvent pas se développer au détriment des citoyens ou des plus petites sociétés enfin une société qui protège, c'est aussi une Europe qui assume des choix clairs en matière de sécurité et défense depuis plus de 2 ans, toute l'Europe est la cible d'attentats sans cesse plus meurtrier, une réponse concertée une protection forte au niveau de l'Union est indispensable, monsieur le ministre, Madame la Ministre, la séquence de questions qui suivra devrait nous permettent d'examiner, nous interroger un petit peu plus en avant sur les actions menées dans ce domaine en matière de défense, l'Europe pourrait aussi se doter d'une force commune d'intervention dans le budget défense commun, telle que l'a proposé le président de la République est telle que nous l'avons retrouvé dans votre intervention Monsieur ministre il y a quelques minutes, nous voulions pas aussi la dimension du renseignement dans la lutte contre le terrorisme, le renseignement se coordonnent s'organisent au niveau européen pour conclure et vous l'aurez compris monsieur le ministre Madame ministre, chers collègues, le groupe Union centriste que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui à cette tribune soutient totalement les démarches entreprises par le président de la République pour refonder l'Europe et lui redonner tout son sens et pour la première fois depuis de nombreuses, en nous avons le sentiment que la France retrouve une place de leader, une parole dans la construction européenne et ce dans un partenariat de bon aloi avec nos voisins allemands oui, chers collègues, nous avons besoin d'Europe et surtout d'une Europe forte qui puisse jouer un rôle de pivot et de stabilisateur, vous avez aussi compris que nous ne partageons pas la vision de mon prédécesseur avait à cette tribune, vision d'assurer spectable mais il faut pas exploiter toutes les facettes d'une volonté de catastrophe ou de décliner séisme déclinistes pardon pour être encore plus explicite : chaque collègue nous sommes fiers de siéger dans cet hémicycle devant le drapeau tricolore mais aussi devant le drapeau de l'Europe. Merci mon cher collègue. La parole est maintenant au président Didier Guillaume pour le groupe socialiste et républicain.

Pas de très nombreuses années, un débat dans cet hémicycle, sur l'avenir de l'Union européenne aurait paru incongru aux parlementaires que que nous sommes tellement il n'y avait pas de débat sur la nécessité de la construction européenne. Nous nous accordions sur la réalité de cet avenir. Nous accordions sur le besoin de cet avenir est presque sur les modalités de cet avenir. Est-ce toujours le cas. La question se pose, et ce débat doit y répondre et vous Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, vous devrez amener avec le gouvernement, ces réponses-là et les apporter au peuple français. Cette sérénité, cette confiance dans le projet européen, nous ont fait oublier la nécessité de l'expliquer et surtout de le penser, voire de le repenser aujourd'hui l'Union européenne vit une crise majeure, une crise comme un an n'a jamais connu auparavant une crise qui peut avoir des issues. La fin de l'idée européenne de l'Europe telle que la bâtir nos prédécesseurs, ce serait un désastre politique et humain, ou alors le redémarrage d'une Europe de prospérité et de solidarité. Et nous devons avoir la volonté chevillée au corps de réinventer le rêve européen oui, Monsieur le Ministre, il faut un sursaut, il faut un cap clair pour une vraie refondation de l'Europe. Au moment où l'euroscepticisme gagne les rangs des Français et plus largement des citoyens européens. L'Union traversent des crises en donnant l'impression d'une totale non maîtrise des événements ou les peuples d'Europe sont de plus en plus méfiants vis-à-vis du projet européen, ce type de débat est utile et devrait même être plus courant. Monsieur lui je veux d'emblée vous assurer de notre soutien pour tout ce qui ira dans le sens d'un renforcement de l'union d'un approfondissement du projet européen et surtout d'une dynamique démocratique européenne. Nous vous soutiendrons parce que notre pays en a besoin parce que vous aurez besoin de la force du Parlement pour vous exprimer pour exprimer une position claire de la France sur la scène européenne parce que nous croyons que c'est dans l'accomplissement d'un projet européen que les peuples d'Europe seront mieux protégés tant termes de sécurité physique que de garanties sociales. Mais sachez que notre exigence et notre vigilance seront fortes et constantes. Nous croyons dans le projet européen parce que nous reconnaissons ce qu'il a apporté aux peuples européens depuis 60 ans, mais aussi parce que nous avons la volonté de corriger les erreurs qui ont pu émaillé sa construction, contrairement à ceux qui ont baissé les bras, nous pensons l'Europe comme un enjeu politique primordial faire table rase, serait une facilité et une erreur historique et quel reniement, quel démission intellectuelle quel déshonneur pour ceux qui veulent aujourd'hui faire disparaître les symboles des Européens comme par exemple le drapeau, c'est absolument inacceptable, le président de la République a dit qu'au Conseil qu'au prochain conseil européen, la France sur une déclaration solennelle pour reconnaître le statut de l'hymne et du drapeau européen, nous y sommes totalement favorable parce que la politique et la construction européenne, c'est aussi une affaire de symboles et bien sûr construire et plus complexe, plus long, plus difficile que de renier mais bien plus utile au peuple, c'est dans cette nouvelle construction européenne que nous souhaitons nous diriger et à ce titre, je souhaite vous alerter sur 2 dangers qui pèsent sur ce projet le 1er est celui du risque de l'éclatement, il a déjà commencé les tenants de l'explosion de l'implosion du projet européen sont nombreuses : notre mobilisation, votre action doivent être totale contre ce risque, nous devons y répondre en affirmant notre volonté d'une Europe intégrée et unie le phénomène britannique n'est pas isolé dans notre pays, la dernière élection présidentielle a montré que la remise en cause de l'Union étaient de plus en plus forte sous 2 formes différentes à l'extrême droite et à l'extrême gauche, les opposants à l'Europe, les eurosceptiques en fait plus de 40 en Allemagne, l'extrême droite est entrée au Parlement Hongrie en Pologne, les opposants au projet européen sont même au pouvoir, la menace donc de l'éclatement de l'Union n'est pas que virtuel et si une partie des Britanniques regrettent déjà leur sortie, personne ne peut dire ce qu'un référendum du même type d'honorer aujourd'hui dans d'autres pays, ce mouvement pourrait devenir une lame de fond contre toute espèce de solidarité, c'est d'ailleurs bien cette volonté de ne pas payer pour les autres, qui a présidé pendant des années au traitement du dossier grec jusqu'à ce que la menace du Brexit fasse évoluer les positions, la France a été à la pointe, il y a joué un rôle déterminant au règlement de la crise grecque, la France compte et doit continuer à compter et à peser dans le concert des nations. Ce danger d'éclatement doit donc nous rappeler au principe de solidarité au sein de l'Union, la construction purement économique à trop écarté ce besoin de solidarité entre les peuples, alors que nos sociétés ont été de plus en plus interdépendant ce paradoxe doit donc être résolu dans une nouvelle phase du projet européen : certes, il faut aller dans le sens d'une union monétaire renforcée d'un budget efficace aux ressources propres de l'harmonisation des politiques, notamment fiscales, vous les avez évoqué, monsieur le Ministre, mais bien, il est absolument indispensable d'aller vers une convergence sociale avec l'adoption d'un socle européen des droits sociaux, sous peine d'un retour en arrière de l'idée européenne par une grande majorité de nos concitoyens. La solidarité, la solidarité européenne, c'est aussi le partage sur les forces de sécurité, la France, d'autant plus avec le départ du Royaume-Uni ne peut plus assumer seul, ou presque, seul, la protection de tout un continent, le contexte terroriste et le besoin du renforcement militaire de notre pays, a montré l'urgence d'une plus grande unité militaire en Europe et je parle devant un expert, les propositions du président de la République en la matière sont fortes, espérons que le projet européen de défense puisse enfin voir le jour le 2ème écueil sur lequel nous serons vigilants et celui de la déconnexion du projet européen, la perte d'espoir dans l'Europe ne vient pas de nulle part parmi les erreurs du passé que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien l'éloignement des citoyens ce que, de ce qu'on appelle la technostructure qui a été la plus terribles de la directive Bolkestein sur les travailleurs détachés de la politique agricole commune à Schengen, les Français sont souvent inquiets et interrogatif l'éloignement a attisé l'exaspération pendant que la crise montrer d'autres failles du projet européen, notamment avec l'absence d'Europe sociale, il n'est plus temps de se satisfaire d'accords entre gouvernement, mais de satisfaire les attentes légitimes des citoyens ne refaisons pas les erreurs du passé n'éloignons pas plus l'Europe des citoyens ne construisons pas de nouvelles instances sans lien démocratique n'empilant pas les institutions comme on parfois si bien le faire, au contraire, Monsieur le Ministre, nous vous demandons de réfléchir constamment tout nouveau projet toute nouvelle institution européenne se fasse avec la volonté de mettre plus de démocratie dans l'Europe. Le Parlement européen doit ainsi obtenir plus de pouvoirs parce qu'il représente la volonté citoyenne, la démocratie, la volonté du peuple, c'est bien le lien entre décision et démocratie qu'il faut renforcer quand nous parlons de projet démocratique, bien avant les débats légitimes sur les modalités d'élection. Nous veillerons à ce que vous preniez ce chemin d'une Europe plus démocratique, là encore vous aurez sûrement des opposants, certains vous expliqueront que ce ne sont que des mots qui ne produiront aucun effet mais croyez-nous, la démocratie n'est pas qu'un mot, elle est un projet en elle-même et l'Europe a besoin de a besoin de ce projet démocratique qui, seule la rapprochera des citoyens démocratie et solidarité, ce sont les 2 principes que nous voulions apporter au nom de notre groupe à ce débat sur l'avenir de l'Union européenne parce que l'Europe doit s'affirmer comme une puissance souveraine, Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué dans votre propos, notre projet européen a besoin d'une boussole d'une identité et ses principes peuvent y contribuer, l'ancrage des symboles européens dans notre pays, participera aussi à la progression du sentiment européen, vous nous trouverez donc avec vous pour contribuer au débat, vous trouverez aussi à vos côtés contre tous ceux qui veulent démanteler l'Europe contre ceux qui prônent le repli, la suppression des symboles au populisme sans limite, répondez par un projet démocratique à la folie démagogique des extrêmes, répondez par l'aspiration à plus de solidarité parce que la France a toujours été du côté des bâtisseurs de notre espace commun parce que la France a un rôle éminent à jouer dans la nouvelle phase qui s'ouvrent, parce que la France avec l'Allemagne demeureront au moteur solide au milieu des autres nations parce que vraisemblablement il faudra un nouveau traité de l'Élysée Monsieur le Ministre, assument ensemble notre volonté européenne inébranlable assumant d'être les fers de lance de sa reconstruction assumant notre histoire assumant quelles qu'en soient les difficultés, il y en aura, quel que soit le travail immense à accomplir, il sera là et quelles que soient les obstacles à lever oui, assumant que nous demeurons des travailleurs infatigables pour continuer à bâtir cette belle idée européenne et que demain encore tous ensemble, nous puissions dire vive l'Euro. Monsieur le président. La parole est maintenant notre collègue. Colette Mélot le groupe République et Territoires les indépendants. Vous avez 6 minutes ma chère collègue. Vous avez la parole. Monsieur le président, Monsieur le ministre madame la ministre, messieurs les présidents de commission chers collègues. Le 25 mars dernier se dérouler les célébrations du 60ème anniversaire du traité de Rome. Un événement propice à dresser le bilan de la construction européenne. De fait, si le projet européen a connu une progression incontestable élargissements successifs, mise en place d'une citoyenneté européenne espace Schengen : création de l'Euro, programme éducatif de nombreux périls le menace le Brexit la montée des populismes la crise Meagher migratoire mais l'Union européenne est une force pour la France et nous devons sortir des clichés sur l'Europe, de nombreux responsables politiques dénonce Bruxelles, oubliant que les États-membres gardait un rôle déterminant dans les prises de décision de l'Union, à titre d'exemple, il dénonce l'échec de Schengen tout en ayant refusé pendant des années de conflit et pleinement aux institutions communautaires le contrôle aux frontières et de donner un budget crédible pour assurer cette mission, nous devons être unis pour être souverain selon la trajectoire prévisionnelle tous les 10 ans, un pays européen sortira du G8 pour conserver une puissance politique majeur et maîtriser notre destin nous devons présenter un franc fort et uni les souverainistes français se trompent de combat en faisant de l'Union européenne, l'adversaire alors qu'il s'agit d'un formidable levier de reconquête de notre souveraineté menacé par nos dettes ou par notre dépendance à certaines matières premières. Nous avons besoin d'une Europe puissance, une Europe qui maîtrise ses frontières qui soit plus cohérente écono qui mi que ment et socialement afin d'éviter des concurrence déloyale entre les États membres, une Europe qui protège son marché intérieur, face à des produits qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos entreprises, à nos agriculteurs enfin une Europe qui doit faire confiance aux territoires en respectant pleinement le principe de subsidiaire sur certains sujets, l'échelle européenne est adéquate sur d'autres, ce sont les États ou les collectivités locales qui sont plus efficaces, reconnaissons cette réalité, le discours du président de la République sur la question européenne va dans le bon sens, il est volontaire évoque plusieurs pistes de réflexion intéressante en termes de souveraineté, d'unité et de démocratie, le gouvernement semble vouloir prendre à bras-le-corps le sujet européen trop souvent laissé aux extrémistes de tous bords et nous saluons cette volonté au sein du groupe Républicains et Territoires les indépendants. Nous partageons par exemple pleinement le projet du président de la République et du gouvernement de donner des outils à l'Union européenne afin de garantir la sécurité à la fois en terme de lutte contre le terrorisme, de défense et de Prozac section civile nous partageant sa détermination de prendre en compte la question migratoire toujours d'actualité, nous approuvons l'idée de faire de l'Union, le leader mondial du développement durable, bien sûr, nous serons extrêmement vigilants sur l'application de ces orientations leur déclinaison en propositions afin que ces mots soient réellement suivis de faits, l'Union européenne ne peut se suffire de mots, il faut des actes l'idée européenne doit être partagée par le plus grand nombre, les citoyens doivent se réapproprier la construction européenne et je profite de ce débat pour soutenir l'idée des conventions démocratiques sur la refondation de l'Union européenne que le président de la République a d'ailleurs évoqué lors de son discours à Athènes, nous devons reconnaître la défiance que certains citoyens français 0 européens ressentent face à la construction européenne, même si son image s'améliore auprès de nos concitoyens, nous ne pouvons ni ignorer ni ni à cette réalité, il est indispensable de communiquer, d'échanger et d'agir pour redonner du souffle et de l'énergie au projet européen trop souvent dans le passé, les responsables politiques ont construit l'Europe sans les citoyens, cela a créé de la défiance de la méfiance, cela entraîne le non au référendum sur le traité constitutionnel en 2005 et pourtant l'Union européenne a engendré de belles réussites, notamment pour la jeunesse, cette année le programme Erasmus fête ses 30 ans, le programme d'échanges universitaires européen rebaptisé Erasmus plus en 2014 et l'un des plus grands et incontestable succès européen depuis 1987 année de sa création, plus de 3 millions d'étudiants ont bénéficié du programme aujourd'hui, ils sont environ 270000 à partir chaque année, confirmant la réussite d'Erasmus plus qui intègre désormais un volet professionnel mais qui reste encore à mon sens trop peu utilisé, il sera utile d'ailleurs que nous abordions cette question lors du débat sur l'apprentissage en conclusion : l'Europe est une nécessité les les enjeux n'ont jamais été aussi fort et c'est la raison pour laquelle il faut associer plus largement encore, les Français, plus que jamais, les Européens doivent se retrouver pour défendre leurs valeurs et renforcer notre économie plus que jamais, les Européens doivent reprendre leur destin en main, pour ne pas devenir, selon les mots de l'ancien commissaire européen, Michel Barnier, je le cite un continent sous influence ou sous-traitants, le Parlement prendra évidemment toute sa place dans les débats à venir, bien sûr, il y a la commission des affaires européennes, notre groupe République et Territoires les indépendances investira également tant cette question est au coeur de notre ADN mais, chers collègues, l'Union européenne est une chance pour la France, nous n'avons pas le droit de la gâcher. Monsieur le ministre madame la ministre, messieurs les présidents de commission chers collègues. quelle Europe pour demain si on vend aujourd'hui à ce qui se joue à l'Espagne, on pourrait se dire : voilà un obstacle de plus au grand projet européen le réveil identitaire qui agissait États membres un voisin, un ami de la France, nous savons qu'travaille aussi d'autres pays. L'entrée massive ou Bouddha, c'est-à-dire de la vidéo aux dernières élections allemandes, a une nouvelle fois démontré le poids croissant des mouvements nationalistes, populistes et eurosceptiques au sein de plusieurs États membres, la France est déjà papa à cette tendance,

terrorisme, l'Europe est sur tous les fronts, avec des résultats, il faut le souligner certains prête beaucoup de mots à l'Union européenne, ça je ai demandé ce que seraient chacune des pays européens, seule, isolée face à la puissance démographique et industriel de la Chine face à l'hégémonie financière américaine ou encore à terme face aux graves régionaux qui s'organise aussi bien à la vie à l'Amérique du Sud, en effet, dans le monde, telle qu'il est aujourd'hui l'addition des forces du nécessité est une condition bien sûr économique, la plupart des États-membres de l'Union européenne, contrairement à ce que certains Anne Reiser croit que c'est devenu la Grèce comme tous les mécanismes de son otage de dérégulation mis à l'oeuvre depuis 2010, quel serait l'état de nos frontières Frontex, l'accord avec Ankara ou bien d'autres instruments venus depuis 2015 contenir un mouvement migratoire avec lequel il faudra vivre. Naturellement, beaucoup reste à faire, mais quelle que soit l'âme vers la tâche : nous ne devons pas attendre d'être au pied du mur pour agir trop souvent certaines outils que j'ai cités sont intervenus dans l'urgence par soi-même, c'est l'émotion qui a accéléré politique, comme ce fut le cas pour pour la politique migratoire parce qu'encore innocent échoué sur une plage avait heurté les consciences, c'est regrettable, attendant malgré celle du village ces retards, l'Union européenne doit demeurer notre MDC qui me horizon la déclaration de Bratislava le je cite l'Europe il ne remplit pas parfaite, certes, mais c'est le meilleur instrument dont nous disposons pour relever de nouveaux défis, le président de la République a rappelé que l'Europe était citation encore une idée portée les plier siècle par les pionniers, les optimistes des visionnaires et que chacun sait ce qu'il nous appartient de nous la réapproprier oui, mes chers collègues, les personnes Nater Andaman de l'Europe, nous avons aujourd'hui le devoir de la réinventer le président a livré sa vision sur l'Europe, une vision fondée sur le concept de souveraineté européenne et pour ma part avec président d'un groupe profondément européenne, je ne peux que me réjouir de cet élan et ce d'autant plus qu'il a été plutôt bien accueillie par nos partenaires, le président les c'était nécessaire souveraineté en matière de défense, le contrôle des frontières, de politique étrangère de transition écologique de numéros de mutation numérique et, bien sûr, de puissance économique et industriel, Rihanna mais oui, dans la plupart des propositions valser, au contraire, et certains d'entre elles assez concrètes sont déjà dans les discussions qui animent régulièrement le Conseil européen d'autres convergent aussi avec le scénario 5 faire beaucoup plus Southam formalisée dans le livre blanc sur l'Europe présenté au début de l'année par Jean-Claude Junker, mais puisqu'une vision pour plus Europe aboutisse, il faut que chacun des États-membres se retrouve sur l'essentiel, que les valeurs que nous partageons soit clairement approuvé la première Londres, là c'est la solidarité, et ce n'est pas une tâche facile que l'encourager davantage, elle a été chaud mis la rue est au cours des dernières années, le Brexit en est un exemple,

aucune convergent du fiscales, sociales ou environnementales ne peut aboutir, homme minimum de bonne volonté partagée mais comment renforcer cette: faut-il arrêter quand elle fait défaut, la réponse doit passer par une réforme destitution, cette question ne doit pas être tabou

qui était momentum politique Marc aussi un jour avoir négocié et signé le traité de Rome contre lesquels Orphée et à me poser à l'administration, sa vision politique mais cette Europe-là n'était pas l'Europe des normes et des règlements et directives qui ne fait plus rêver personne,

La parole est à Monsieur André Rey charter pour le groupe Les Républicains pour 15 minutes.

C'est le président, messieurs les présidents, madame la ministre mis chers collègues, il y a encore peu de temps, le fait même d'évoquer l'avenir de l'Union européenne pouvait apparaître comme la marque d'un optimisme un optimisme forcené dans celle-ci semblait à bout de souffle depuis plus de 10 ans, elle a en effet vu se succéder les anus horribilis comme on a dit chacune charriant son lot de crises nouvelles certaines plus violente que les autres ont fait vaciller sur ses fondations notre notre édifice commun et ont transformé les dirigeants européens ont pompiers contraints de combattre les uns après les autres les incendies qui menaçaient de tout ont porté, même si le feu couve toujours sous la cendre, le tumulte de ces années noires semblent aujourd'hui pour un temps au moins derrière nous et il est à nouveau permis d'envisager un avenir pour l'Union européenne au travers de ses discours d'Athènes et de la Sorbonne, c'est ce à quoi s'est employé, le président de la après un quinquennat marqué malheureusement par un effacement, fort de la France sur la scène européenne, cette expression était plus que nécessaire pour remplacer notre pays au centre du jeu. Et de fait, sur ce point au moins monsieur Emmanuel Macron a réussi son pari, puisque les propositions françaises alimente largement le débat sur ce qu'il est désormais convenu d'appeler la refondation de l'Europe, cela veut-il dire pour autant que le cadre proposé par le chef de l'État fasse consensus à l'évidence, la réponse est non. Les constats qui se sont pourtant bien lucide face aux grands défis contemporains, l'Europe et le cadre naturel de notre action collective oui trop longtemps la construction européenne s'est fait à l'abri des peuples sans qu'il n'ait réellement de prise sur elle, oui les élargissements qu'a connu l'Europe ont accru sa diversité Andante inévitable une plus grande différenciation dans notre coopération. Mais même si nous partageons un certain nombres de ses préconisations le projet présenté par le président de la République nous laisse perplexe en 1er lieu parce que même s'il s'en défend il s'agit bel et bien un mouvement vers une Europe fédérale, qui nous est proposé pour une avant-garde, dont la France aurait semble-t-il vocation à prendre la tête, sinon comment comprendre les innombrables références faites à la souveraineté européenne cette souveraineté qualifiée de réelles qui semble renvoyer au rang de fiction, la souveraineté nationale si on au soir du 7 mai les Français ont clairement rejeté la voie menant au démantèlement de l'Union européenne, ils n'ont pas pour autant plébiscité cette Europe fédérale qui apparaît comme l'horizon tracée par monsieur le président de la République, certes, nous sommes tous conscients de l'existence d'une seule et même civilisation rassemblant les peuples européens dans une identité qui leur est propre et qui les distinguent du reste du monde. Mais chercher à forcer leur destin fédéral, c'est perdre de vue que leur évidente proximité n'efface pas leur diversité, ce n'est pas en multipliant les instances supranationales que l'Europe sera nécessairement plus efficaces ou mieux accepté son salut ne réside pas forcément dans la mutualisation systématique mais plutôt dans ce que nous appelons, nous, une articulation intelligente des principes de solidarité et de responsabilité au service d'objectifs communs, bien plus que d'un projet institutionnel fédéral cette avant tout d'un projet politique de civilisation de notre continent aujourd'hui besoin, c'est même plus que jamais mais, chers collègues, sa principale raison d'être face aux mutations et aux convulsions du monde contemporain, pour cela, il y a tout d'abord indispensable d'ancrer l'Europe dans un territoire qui reflète son histoire et son identité des frontières stable et cohérente, sont une condition essentielle pour que les Européens prennent davantage conscience de même l'incertitude géographique devenu symbole de l'Ain définition politique ne leur permet pas d'appréhender la nature de leur projet commun. De la mer Baltique à la mer Égée, nous croyons que les frontières de l'Union doivent être stables en conséquence, nous devons nous devons avoir le courage de clarifier dès maintenant la nature de nos rêves, notre relation avec nos voisins, cela impose en particulier des trop clair quant à la poursuite ou non. Du processus d'adhésion de la Turquie, dont Jean-Claude du maire lui-même estimait récemment qu'elle s'éloignait de l'Europe à pas de géant, il faut en tenir compte plusieurs États-membres d'ores et déjà réclamé cette clarification, il faut désormais passer aux actes, la 2ème priorité réside, selon nous, dans la nécessité de trouver une plus juste articulation entre construction européenne et expression des démocraties nationales car le fait national, celui des peuples et des États reste, selon nous, le creuset fondamental de la souveraineté de la légitimité politique et donc de l'exercice de la démocratie personne Madame la ministre ne s'oppose naturellement à l'organisation 2018 2 conventions démocratiques qui peuvent s'avérer fort utile, mais je crois qu'il faut avant tout renforcer le rôle tenu par les parlements nationaux rapprocher l'Europe des citoyens restera un voeu pieux, s'ils ne sont pas en mesure d'agir concrètement sur le débat et le processus législatif, il me semble, alors difficile de soutenir l'élection d'une moitié, a-t-on dit, aujourd'hui, on a plus parlé de moitié du Parlement européen sur des listes transnationales, sauf à vouloir éloigner encore plus les élus de leurs électeurs, au contraire, un pouvoir d'initiative devrait être donnée aux parlements nationaux pour leur permettre de contribuer positivement à l'élaboration des législations européennes, ce droit d'initiative devrait d'ailleurs aller de Pair avec l'instauration d'un droit de véto, leur conférant la capacité certes sous certaines conditions, de stopper l'examen d'une proposition législative qui ne nous convient pas, nous devons également nous interroger sur la répartition des compétences entre l'Union et les États, l'Union européenne doit définir sa valeur ajoutée par rapport à leur action, cela passe nécessairement et notamment par un réel examen en profondeur du Champ des compétences partagées, car il faut savoir et pouvoir mieux expliquer qui fait quoi en Europe, sans attendre la conclusion de ce travail, l'Union doit se concentrer sur un socle commun constitué de ses compétence exclusive du marché unique et des secteurs fondamentaux pour sa compétitivité et sa stabilité future comme par exemple la défense les frontières extérieures, la recherche, le numérique, l'énergie, les grandes infrastructures de transport, de transport et de communication ou encore bien sûr la lutte contre l'optimisation et l'évasion fiscale, nous avons par ailleurs laissé se développer en Europe, une Europe de l'accessoire, il faut s'en détourner, car l'Union n'a pas été fait pour réagir régenter les détails de notre vie quotidienne, elle a été faite pour permettre d'élaborer collectivement des réponses aux enjeux d'envergure continental, la simplification législative à l'oeuvre dans la plupart des États-membres, doit devenir la norme

apparaissent aujourd'hui comme une impasse qui doit céder le pas à l'exercice en commun de compétences par un cercle restreint de pays volontaires capable et responsable, notre objectif n'est pas la constitution d'un hypothétique noyau dur en pointe dans tous les domaines, la France travailleurs pas automatiquement vocation à prétendre faire à chaque fois, partie d'un peloton de tête des plus allant, il ne s'agit pas non plus de déconstruire l'acquis communautaire en proposant une Europe à la carte sur tous les sujets, car sinon on finira par être une Europe à 27 vitesses, il s'agit plutôt d'accepter que la différenciation désormais le chemin le plus praticable pour toute initiative nouvelle d'importance, or les compères à ce les coopérations renforcées sont trop souvent trop difficiles à rassembler et les règles en la matière sont faites pour ne pas marcher assurément procédure d'activation doit donc être considérablement assouplis. Mais le 3ème chemin arpenté pour bâtir l'Europe du XXIe siècle, et celui de la protection dont on a beaucoup parlé d'ores et déjà, l'Union européenne n'aura de sens aux yeux des comptes des citoyens que si elle se montre capable de mieux les protéger. Premières de la protection des frontières, l'exigence de contrôle de notre espace n'a jamais été aussi forte, nous devons donc assurer la pleine maîtrise de nos frontières extérieures, la montée en puissance du corps européen de gardes-côtes de garde-frontières est à ce titre, indispensable, je reste toutefois attaché au fait que son intervention reste conditionné à l'accord des États membres concernés je ne souscris donc pas à l'idée de créer une police européenne des frontières dont l'intitulé, laisse à penser qu'elle pourrait agir de manière indépendante sur les territoires nationaux le développement hotspot devra par ailleurs être accélérées et surtout les personnes ne bénéficiant pas du droit d'asile devront être éloignés systématiquement cela sous-entend néanmoins que les pays d'origine, accepte de l'aéroport reprendre sur le territoire et c'est la raison pour laquelle la coopération avec les pays tiers et notamment l'aide financière qui qui leur est octroyé devrait être conditionnée à la signature et à l'application effective d'accords de réadmission 2ème axe de cette protection, la défense, les Européens hésitent encore à regarder en face la réalité d'un monde qui n'est plus seulement instable mais dangereux, ils doivent pourtant d'urgence recouvrer l'autonomie stratégique qu'ils ont délégué aux États-Unis, cela ne signifie pas la constitution d'une armée européenne dans les conditions de création ne seront peut-être jamais réunie, ça ne signifie pas non plus la fin de notre alliance avec les États-Unis, notre ambition doit être selon nous de rééquilibrer la coopération euro-Atlantique en rapprochant en Europe nous vision stratégique globale et en renforçant le niveau et la cohérence de nos moyens financiers capacitaire et opérationnel, les récentes initiatives en la matière, vont dans le bon sens, assurément, elle pourrait être utilement complété par un semestre européen de la défense, destiné à améliorer notre coordination stratégique assurer la montée en puissance de nos engagements financiers. Et entamer un développement concerté de nos capacités, mais il faut également consolider notre politique industrielle de défense, à ce titre, nous devons développer des programmes communs d'armement pour améliorer l'interrompent opérabilité armées accroître le volume de la commande publique et inciter les industriels à procéder au rapprochement nécessaire pour y répond : cela nécessite d'ouvrir davantage les marchés défense au niveau national, mais pour donner un sens à cette ouverture, il nécessaire d'appliquer à ces marchés particuliers la préférence communautaire, abandonnés dans les autres domaines du marché intérieur 3ème axe de la protection de renforcement de la zone Euro depuis le déclenchement de la crise, celle-ci, la zone Euro s'est doté de règles plus robuste et de nouveaux outils pour assurer sa viabilité, sa résilience. Mais les traces laissées par la crise sont encore profondes et ont miné la confiance entre les États-membres. Les solutions qui appelle à un nouveau partage des risques comme l'émission commune de dette publique ou la création d'un budget de la zone Euro destiné à organiser une union de transferts ou à amortir les chocs via par exemple une assurance chômage européennes ne peuvent recueillir notre assentiment ni d'ailleurs celui de nombre de nos partenaires, c'était avant tout dans les États membres, que se joue l'avenir de la zone Euro, car c'est de leur responsabilité individuelle que dépend sa cohérence, nous devons donc au contraire nous concentrer sur la réduction des risques. Cela passe néanmoins effectivement par le renforcement du Cadre de gouvernance, nous sommes d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de créer une fonction de coordinateur de la zone Euro mais qui selon nous serait avant tout chargée d'assurer une meilleure coordination des politiques économiques et une surveillance budgétaire renforcée, il est parallèlement nécessaire de progresser sur la voie de la convergence fiscale mais également sociale, on l'a dit avant moi, s'ils sont l'expression des choix collectifs souverain fait par les peuples européens les différentiels de fiscalité, d'orientations de politique sociale, mais des pratiques de dumping qui mine l'efficacité du marché unique et de la zone Euro, ainsi que la confiance entre Européens, la convergence va donc s'esquisser sans attendre en 1er lieu la solidarité qui prévaut dans la zone Euro, il y a le mécanisme européen de stabilité ne peut aller sans responsabilité en matière fiscale, on ne peut imaginer qu'un pays puisse bénéficier de la garantie de ses partenaires, tout en poursuivant une politique de concurrence fiscale qui, en réduisant la croissance dans les autres pays de la zone Euro contribue à y créer creuser les déficits et dégradé le marché du travail, sans procéder à une uniformisation complète cette convergence pourrait s'appuyer sur un rapprochement du fonctionnement global des systèmes nationaux et surtout sur un dispositif de serpent serpent fiscal et social encadrant à tout le moins, certains taux d'imposition ou le niveau de certaines prestations sociales, le développement d'une collaboration étroite avec l'Allemagne serait effectivement un bon point départ Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avait ouvert la voie en 2012 avec un livre Vert sur les points de convergence franco-allemand sur la fiscalité des entreprises, cette dynamique doit être relancée 4ème axe de la protection, la défense de nos intérêts dans la mondialisation, nous souhaitons mettre en place des mécanismes raisonné de protection de notre économie, l'Euro, l'Europe offre à ses partenaires, qui sont également ses concurrents un accès quasi totale à ces marchés alors que même n'ont aucune hésitation à protéger le nord, dans le pire des cas, certains d'entre eux pratiquent une concurrence ouvertement déloyale ou le dumping, voire la contrefaçon est érigée en modèle économique, c'est inacceptable, notre continent doit démontrer qu'il est désormais prêt à défendre sans complexe ses intérêts la conclusion des accords commerciaux devraient en 1er lieu être réellement soumise au principe de réciprocité pour protéger son modèle Europe devrait par ailleurs mettre en place des taxes anti-dumping contre les biens, services et capitaux ne respectant pas les normes internationales de base et adopter des sanctions fermes à l'encontre des pays contrefaisant massivement des produits européens, affirmer l'identité de l'Europe, mieux articuler action européenne et démocratie nationale et apporter plus de protection aux Européens, voilà, Madame la Ministre, mes chers collègues, brossé à grands traits quelques pistes d'évolution qui nous permettront de Renault et du sens à notre coopération et d'emporter assurément l'adhésion de ses concitoyens, je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à monsieur Jean Bizet et président de la commission des affaires européennes pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre chargé des Affaires européennes, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je me félicite de cette occasion de débattre avec le gouvernement de l'avenir de l'Union européenne, le Sénat avait en quelque sorte pris les devants, il y a quelque temps déjà, à la demande du président Gérard Larcher nous avions avec Jean-Pierre Raffarin crée un groupe de suivi du Brexit et de la refondation de l'Union européenne, un groupe commun aux commissions des Affaires européennes et des Affaires étrangères, retrouver l'esprit de Rome : telle était l'intitulé de ce rapport est le défi qu'il nous impose désormais de relever au terme de 8 mois de travaux quelques constats à quel constat sommes-nous arrivés la construction européenne est un grand projet et l'Europe est confrontée à de graves crises internes la décision britannique a constitué un choc, c'est un non-sens géostratégiques, gardons-nous d'ailleurs d'encourager les autres forces centrifuges à l'oeuvre, profiterait de l'occasion pour saluer le travail de notre collègue Michel Barnier, qui, avec beaucoup de fermeté et de rationalité, par rapport à l'incohérence et l'inconstance britannique mène l'ensemble des négociations, nous voulons avec le Royaume-Uni une séparation ordonnée la construction d'une relation solide pour l'avenir. Mais un échec des négociations est toujours possible, l'Union doit maintenir sa position, elle est claire, pas de passage à la seconde phase sur les relations futures avant le règlement des 3 questions-clés que constituent la situation des citoyens européens installés au Royaume-Uni, le règlement financier et la question de l'Irlande, monsieur le ministre des Affaires européennes et des forces armées, l'a rappelé tout à l'heure, l'Europe paie aussi son impuissance face à la crise économique et financière aux attaques terroristes et aux chocs migratoires. Pour relever ces défis, une vision et un Leadership font défaut, les États membres ont refusé de s'approprier véritablement le projet européen avec une fâcheuse propension à reporter sur l'Union, la responsabilité de tous les maux, pour s'approprier les seules réussites, nous en avons payé le prix fort, avec une dérive bureaucratique, doublé d'un déficit avec une dérive bureaucratique, doublé d'un déficit démocratique déficit qui a alimenté la montée précisément du populisme, la défiance à remplacer la confiance, il y a en réalité qu'une alternative : soit le sursaut européen soit malheureusement la sortie de l'histoire, le Brexit doit doit précisément donné le signal du sursaut, l'Europe ne doit pas être seulement une Europe espace centrée sur le marché intérieur mais plutôt une Europe puissance assumant véritablement sa dimension politique, le projet européen doit être refondée sur une heure, une vision assumé, porté par les États nations à partir de quelques priorités pour lesquelles la plus-Value européenne est clairement identifié par l'les l'Europe doit se réaffirmer comme puissance, elle doit exercer ses responsabilités en matière de défense dans la lutte contre le terrorisme, la sécurité intérieure et consolider sa réponse à la crise migratoire c'est une attente forte des peuples européens, il faut y répondre : premières puissances commerciales avec la force de son marché unique, on aurait tort de l'oublier, l'Union doit se faire respecter dans les négociations commerciales internationales, ça été rappelé tout à l'heure par notre collègue André Richard, l'Europe doit définir des priorités économiques, à l'image d'Airbus ou d'Ariane hier, elle doit lancer de nouvelles actions pour la croissance et non le numérique, l'énergie sont des priorités : l'Europe doit aussi aller vers la convergence fiscale, la politique de la concurrence doit être mise au service de la reconquête industrielle et de l'emploi et non plus continuer constituer une entrave à l'émergence de champions. Européen, l'Union européenne doit parachever la gouvernance de l'Euro, avec un contrôle démocratique effectif impliquant pleinement les parlements nationaux. S'agit. également de renforcer la cohésion européenne en progressant vers la convergence sociale le dossier des travailleurs détachés en soulignent l'impérieuse nécessité. Et puis aussi en modernisant la politique de cohésion, cette politique est nécessaire aux pays d'Europe centrale et orientale qui ont rejoint l'Europe mais les obligations qui sont les nôtres en la matière n'a d'égal que leur propre obligation de respecter les valeurs de l'Union, je veux aussi insister sur l'enjeu crucial de la prochaine réforme de la politique agricole commune, nous y avons travaillé avec la commission des affaires économiques et dans sa résolution, le Sénat rappelle la légitimité d'une politique agricole commune, par simple et lisible, il affirme l'importance de la PAC pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de l'Europe toute entière cette Europe recentrée doit respecter pleinement la subsidiarité, elle doit être plus visible, plus proche des citoyens, elle doit faire toute sa place aux parlements nationaux le fonctionnement institutionnel doit être revue avec notamment une diminution du nombre de commissaires, l'Europe a également besoin de simplification et de transparence, ceci doit être une priorité permanente, cette nouvelle ambition doit être porté par le moteur franco-allemand, lui seul peut rêver. L'Europe, je dois dire que l'Allemagne cherche des partenaires fiables et fort partenaires: la France, les depuis le 1er jour fiable fort, elle ne pourrait l'être davantage si elle assumer et entreprenez des réformes sans cesse penser toujours repoussé. La relation franco-allemande ne doit pas être exclusive, elle n'en est pas moins décisive, une feuille de route franco-allemande, tourné vers les enjeux du XXIe siècle, telle que la digitalisation de notre économie, donnera une impulsion nouvelle au projet européen. Le pragmatisme conduit aussi encourager le recours aux coopérations renforcées entre les États-membres États-membres volontaires pour avancer, nous l'avons utilisé que trop souvent, je dois le déplorer et à chaque fois que nous l'avons fait nous avons eu du succès, je me rappelle le dernier ou l'avant-dernier en date, qui fut la coopération renforcée sur le brevet communautaire qui a été un vrai succès. Pour dynamiser l'économie européenne, l'Union européenne doit enfin redevenir le projet partagé des citoyens européens, mobilisons les jeunes autour de ce projet Erasmus constitue une formidable réussite, plus de 3 millions du tout. Il y en ont bénéficié, Colette Mélot l'a rappelé tout à l'heure, il faut désormais aller plus loin et mettre en place un Erasmus pour les apprentis, autant de sujets et de dossiers qui nous attend, je vous remercie. Monsieur Christian Courbon, président de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour 8 minutes. minutes. La Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités, bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe, mais ça n'aboutit à rien, il faut prendre les choses comme elles sont, cette célèbre saillie du général De Gaulle nous rappelle à la réalité, la vision de l'Union européenne que nous a livré le président de la République dessine à l'évidence un bel idéal, un idéal élevé qu'il ne peut que résonner dans le coeur des européens convaincus que nous sommes tous bien évidemment mais un idéal qui nous sommes parfois loin très loin de la réalité que nous vivons. La sécurité et la défense en fournissent un bel exemple de saisie, nous profitons pourtant d'un exceptionnel alignement des planètes l'opinion dans la crainte d'une montée du terrorisme à nos frontières est en attente d'initiatives fortes, ça n'a pas toujours été le cas, la Commission européenne a pris des positions inédite dans ce domaine de la défense et les déclarations de la nouvelle administration américaine en faveur d'un pilier européen robuste de l'Alliance Atlantique et qui se prendre en main tout ceci irait plutôt dans le bon sens, prenons garde néanmoins de ne pas susciter des attentes trop peu élevé qui serait forcément déçu. Alors même que le danger est à nos portes, nous le savons bien la défense de l'Europe, c'est-à-dire la défense du continent européen assumé collectivement par nous-mêmes, par les Européens, ce n'est pas pour demain, et disons-le tout Net, ce n'est même pas pour après-demain, alors bien sûr, cela ne doit pas empêcher la France d'être un moteur car il y a aujourd'hui une conjonction astrale jamais observée jusqu'alors il convient d'en profiter, la France est évidemment le pays membres de l'Union européenne le mieux à même de porter la vision politique d'une Europe de la défense, nous qui avons la 1ère armée en Europe, nous qui avons cette culture de l'indépendance stratégique et qui avons toujours pensé la politique européenne de défense, comme un complément de l'Otan. Des avancées importantes sont là aujourd'hui, avec la coopération structurée permanente et le fonds européen de défense, cette coopération structurée permanente issu du traité de Lisbonne a fait des progrès, auquel la France et l'Allemagne sont loin d'être étrangère le conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 13 juillet laissent espérer des résultats opérationnels avant la fin même de cette année dans une démarche inclusive que le Sénat a toujours soutenu, de même le Fonds européen de défense se mettent en place, c'est le cas du volet de recherche depuis avril 2017 avec le lancement de l'action préparatoire et le volet capacité amorcée par l'annonce de la création en juin dernier, d'un programme européen de développement de l'industrie de défense programme pilote pour la prévenir pour la période 2019, 2020, qui vise à soutenir les programmes capacitaire collaboratif à hauteur de 500 millions d'euros par an pour les 2 premières années et la possibilité de monter à un 1000000000 d'euros pour les années suivantes, nombre d'obstacles demeurent pour sa concrétisation pour la période 2010 2021 2017, 2021, il faudra bien sûr passer les élections européennes de juin 2019, il faudra que se mette en place une nouvelle commission européenne qui reprendra à son compte cette belle ambition, dans le cadre d'un budget dont on peut imaginer qu'il sera en contraction, il faudra aussi trouver une future majorité qualifiée au Parlement européen, sur des sujets qui ne vont pas de soi pour de nombreux députés européens mais l'Europe de la défense doit également reposer sur un pilier capacité, c'est-à-dire sur des projets concrets d'équipements mené en coopération industrielle et financière avec nos partenaires membres de l'Union. Ces projets ont bien sûr vocation à recevoir le soutien du nouveau fonds européens de la défense en cours de mise en place, je viens de l'évoquer, l'enjeu est non seulement de rendre crédible l'avenir de notre défense commune, mais aussi d'entretenir et de développer notre base industrielle et technologique en la matière, gage d'autonomie stratégique et à la fois le développement économique, il serait bien que les Européens prennent l'habitude par exemple de concevoir, de développer et d'acheter des équipements militaires issus de l'industrie européenne l'exemple d'un récent marché d'hélicoptères en Pologne, montrent qu'il y a encore quelques marges de progression de ce point de vue, je donne acte au gouvernement des récentes initiatives importantes prises par la coopération franco- allemande, en particulier le programme Euro drônes le prochain standard de l'hélicoptère Tigre, les nouvelles générations de systèmes de combat terrestre et de patrouille maritime ou encore l'espace et la cyber défense il faut encore saluer ici la consolidation du secteur de l'armement terrestre avec le groupe NDS les initiatives décidées le mois dernier avec l'Italie dans le domaine des missiles ou du spatial notamment constitue là encore un bon signal, on reste toutefois en attente des résultats que pourra produire l'accord de principe trouver à l'occasion du déblocage du dossier STX sur la perspective d'un partenariat structurant dans le secteur Naval entre Naval groupe Efic entière nombre de défis industriels et stratégique reste à l'évidence, a relevé Madame la Ministre, tout ceci n'est pas rien, mais nous sommes encore bien loin de pouvoir doter l'Union européenne d'après les mots du président de la République, je cite, d'une force commune d'intervention d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir car, en vérité, chacun le sait bien, la politique d'emploi des forces qui est celle de la France, sa capacité de projection en opération au-delà de ses frontières est une singularité dans l'Union, au Sahel, c'est bien la sécurité des Européens dans leur entier au flanc sud de l'union que nous les Français nous assurons le seul État membre qui partageait notre culture stratégique, le royaume du le Royaume-Uni est en passe de nous quitter et je veux dire ici notre souhait que le partenariat fort qui nous lie dans la défense avec les accords de Lancaster House soit poursuivi et approfondi, la France a une responsabilité particulière pour arrimer les Britanniques à la sécurité du continent européen, les propositions du gouvernement de Madame Theresa May sur le partenariat sans conditions avec l'Union européenne en matière de sécurité et de défense sont certes très encourageante mais mes chers collègues, quel paradoxe : les Britanniques vont garder l'Europe politique, celle qu'ils ont tant décrié, quand ils étaient au sein de l'Union européenne, alors qu'ils ont quitté le marché unique, alors Madame la Ministre, pour conclure sur une note positive, je voudrais me féliciter que la refondation du projet européen soit au coeur des priorités du président de la République et du gouvernement, le groupe de suivi du Sénat sur le Brexit que vient d'évoquer mon collègue Jean Bizet a diagnostiqué le fort risque des constructeurs pour l'Union européenne, de la sortie du Royaume-Uni la diffraction de l'Europe est un non-sens géostratégique à l'heure des pays continents et aura des conséquences lourdes si on ne relance pas le projet européen, la commission des Affaires étrangères de la défense, vous rejoint sur ce point, la priorité, c'est évidemment l'avenir de l'Union à 27 je vous remercie. La parole est à monsieur Vincent et président de la commission des finances pour lui minutes aussi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en septembre, le président de la République et le président de la Commission européenne ont chacun lancé un appel en faveur d'une Union européenne plus forte, or une Union plus forte. Ainsi que l'a exprimé monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une Europe qui soit une véritable puissance économique et financière, une Union plus forte suppose une union économique, monétaire et financière plus forte le Brexit nous pousse à faire de l'Europe continentale, un centre financier majeur, pouvant s'appuyer sur une union des marchés de capitaux, la France doit tirer son épingle du jeu dans la réorganisation en cours et il est positif que le gouvernement ne remettent pas en cause les mesures prises par son prédécesseur pour améliorer la compétitivité de la place de Paris et même reprend dans la loi de finance des mesures proposées par la commission des finances du Sénat, et son rapporteur général, notre collègue de Montgolfier l'avenir de l'Union suppose également de consolider la zone Euro, de nombreuses mesures ont été adoptées ces 10 dernières années pour répondre aux situations d'urgence lors de la crise aujourd'hui le débat sur l'avenir de la zone Euro, être intense mais surtout institutionnels les propositions pas ministre des pas ministre des Finances de la zone Euro budget propre fonds monétaire européen 13 de la zone Euro parlements de la zone Euro, il s'agit là de sujets importants et qui soulève des questions juridiques comme l'anti-illustrer les auditions que nous avons organisé sur ce sujet, en juillet, mais ce débat institutionnel ne doit pas nous éloigner de la question essentielle : la zone Euro serait-elle aujourd'hui en mesure de faire face à une nouvelle crise d'une ampleur comparable ou supérieure à celle de 2008 et parmi les réformes proposées, lesquels sont les mieux à même de protéger les citoyens européens, l'architecture et le fonctionnement de la zone Euro demeurent vulnérables si les mesures, la Banque centrale européenne sont et efficace, les gouvernements ne pourront pas se reposer indéfiniment sur son action. La décision du peuple britannique de sortir de l'Union européenne et les négociations sur le Brexit ne doivent pas nous conduire à remettre à plus tard la réforme de la zone Euro, au contraire, il s'agit d'une raison supplémentaire pour avancer rapidement. à cet égard, 4 ensembles de mesures revêtent une importance particulière pour l'avenir de l'Union économique et monétaire, premièrement avec l'union bancaire et la prise en charge des risques rencontrés par les systèmes bancaires nationaux, nous vivons un test grandeur nature de la capacité des États à gérer ensemble les risques en partageant leur souveraineté, le test n'est pas encore conclure puisque les discussions sur le mécanisme européen de garantie des dépôts bancaires et le fonds de résolution unique sont bloquées et vous nous direz si vous pensez que la nouvelle feuille de route, présentée par la Commission européenne sera de nature à faire avancer les choses, deuxièmement, le mécanisme européen de stabilité doit être renforcé pour répondre aux crises pouvant affecter la stabilité de la zone Euro mais il ne pourra pas devenir un véritable fonds monétaire européen prêteur en dernier ressort des États-membres sans une réflexion préalable sur son contrôle démocratique par les parlements nationaux. Troisièmement, il manque aujourd'hui un mécanisme de stabilisation budgétaire en cas de choc macroéconomique affectant la zone Euro, notamment dans des circonstances où la politique monétaire atteindrait ses limites. Que ce mécanisme prenne la forme d'un budget d'investissement de la zone Euro ou d'une ligne budgétaire dédiée à la zone Euro au sein du budget de l'Union, sa mise en oeuvre, on aura des conséquences sur nos systèmes fiscaux en partageant les ressources en enlevant de nouvelles, là encore, nous touchons à l'essence de la souveraineté des États. à ce sujet, la proposition du président de la Commission européenne d'introduire le vote à la majorité qualifiée, en matière de fiscalité soulève une question cruciale alors que la concurrence fiscale ça tease quels États seraient prêts à renoncer à leur droit de véto sur la fiscalité, la réussite de plusieurs chantiers ambitieux initié par la Commission européenne dépend de la réponse à cette question, enfin la définition d'une politique économique européenne et un pilotage cohérent au niveau de la zone Euro suppose une plus grande convergence des économies des États-membres, les règles de surveillance budgétaire sont particulièrement complexe et sujette à interprétation, le débat actuel sur la flexibilité du pacte de stabilité et de croissance, en est un exemple éloquent à minima une clarification des règles de surveillance budgétaire et de leurs objectif serait donc la bienvenue. S'agissant des réformes structurelles, les recommandations adressées chaque année aux États-membres par leurs pairs, réunis au sein du Conseil ne deviennent pas des éléments des débats publics nationaux la procédure être hors sol elle manque probablement d'ancrage démocratique là encore dans les institutions nationales, la ministre, mes chers collègues, en définitif, la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour rendre la zone Euro plus solide suppose une volonté politique forte et une confiance mutuelle entre membres pour reprendre les mots de Jean Monnet, il n'y a pas d'idée prématurée, il y a des moments opportuns, qu'il faut savoir attendre. Près de 10 ans après le déclenchement de la crise économique et financière, et alors que le Conseil européen est appelée à statuer sur l'avenir de l'Union d'ici mars 2019, le moment est certainement venu d'agir. Pour répondre aux orateurs, la parole est à madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier pour ce débat qui a parmi une expression à la fois complète et marqué presque toujours de cette sagesse qui caractérisent vos travaux. J'appuie la suggestion du sénateur Gattolin de faire de ce débat, un rendez-vous annuel et je sais pouvoir parler aussi au nom de Jean-Yves Le Drian. Je vais revenir sur certains sujets que vous avez soulevé, je crains de ne pouvoir tout traiter dans le temps qui m'est imparti et je resterai évidemment à la disposition des membres du Sénat, comme je le suis depuis ma nomination, et tout particulièrement, quoi que, sans exclusive, ceux la commission des affaires européennes, donc je veux saluer ici l'implication et le travail. Mesdames et messieurs les sénateurs, certains d'entre vous ont exprimé sur l'Union européenne, comme elle fonctionne ou comme les autorités françaises souhaiterait qu'elle soit refondée des encouragements parfois des critiques, soyez-en remercié dans les 2 cas, car certaines critiques sont à l'évidence légitime. Oui, l'Union européenne aujourd'hui et parfois trop bureaucratique et trop peu démocratique, Monsieur Guillaume, vous avez raison, ces critiques doivent être entendus et pris en compte dans les efforts que nous déployons pour une refondation ambitieuse de l'Europe, en revanche, je voudrais réaffirmer avec force que le gouvernement a fait le choix de porter, comme l'a fait le président de la République, une ambition forte pour l'Europe, car c'est en refondant l'Europe que nous retrouverons en la partageant notre pleine souveraineté. à l'échelle de l'Europe que nous serons les mieux armés pour relever les défis d'émigration des mutations technologiques du dérèglement climatique, du terrorisme, nous ne pourront pleinement protéger nos industries et nos employes de ce qui fausse les règles du jeu du commerce international, qu'il s'agisse des biens ou des investissements. C'est par une convergence renforcée par le haut de nos économies. Notamment mais pas seulement au sein de la zone Euro, donc vous avez justement appelé de vos voeux la nécessaire réforme monsieur le Président, et que nous tirons pleinement profit du marché unique, soyez assurés que nous défendrons l'agenda de protection que nous avons exposé à nos partenaires, le gouvernement est pleinement mobilisée pour modifier la directive sur les travailleurs détachés et la partie du règlement sur la sécurité sociale qui en traite les négociations sont en cours pour empêcher des fraudes et le dumping social, nous sommes aujourd'hui en situation d'empêcher l'adoption de textes insuffisamment ambitieux, nous travaillons maintenant à rassembler une majorité qualifiée Monsieur puisque l'unanimité qui est sans doute hors d'atteinte, n'est pas nécessaire, les ministres du Travail essaieront de parvenir à un accord au Conseil du 23 octobre soyez, en tout cas assuré de la détermination du gouvernement j'ai évoqué ces sujets en Pologne, la semaine dernière, je le ferais à nouveau dès demain en Hongrie. Jean-Yves Le Drian, vous a présenté des lignes de force du discours du président de la République à la Sorbonne le 26 septembre une dynamique s'est mise en place, un élan comme là, vous l'avez qualifié Monsieur Ruquier l'appel lancé par le président de la République a eu un écho très important dans les opinions publiques comme auprès des membres du Conseil européen qui l'a rencontré, le 28 septembre, nous devons faire vivre et ont conservé l'ambition, rien ne serait pire que de nous contenter d'un catalogue de mesure qui tendrait à se réduire progressivement, c'est pour cela qu'il était essentiel Katalin les chefs d'État et de gouvernement s'accordent sur la nécessité de refonder l'Europe ce qu'ils ont fait, c'est pour cela que nous devions démontrer que ça gêne, ce n'était pas une préoccupation française mais une cause européenne le fait que le président du Conseil européen, monsieur, tout ce qui était mandaté pour présenter dans les prochains jours une feuille de route européenne qui a vocation à partager notre vision est fondamentale et répond à ceux qui, essayer d'opposer notre approche et l'approche communautaire Donald ce qui était d'ailleurs à Paris ce midi pour en débattre avec le président de la République.

Mais cette méthode fait aussi toute sa place au dialogue avec tous nos partenaires, bien entendu, d'abord avec l'Allemagne oui, nos hommes objectifs sont ambitieux, y compris dans le domaine de la défense Monsieur le Président, quand bon hé oui, sans doute il ne auront pourront pas tous être atteints, tout de suite à 27. Ceux qui veulent aller plus loin, plus vite doivent pouvoir le faire sans être empêchés, mais les travaux que nous préparons sont ouverts à tous, avec pour seul critère un niveau d'ambition partagée, tous les États qui adhère à cette volonté, pourront participer au groupe de la refondation européenne avec, bien entendu, les institutions européennes d'ici l'été 2018, ce groupe travaillera pour préciser et proposer des mesures qui traduiront concrètement cette ambition. Il devra notamment déterminer pour chaque politique et sans tabou, compte tenu des percées qu'un nombre significatif d'États envisage, s'il est possible d'avancer à 27 c'est un changement de traité est nécessaire, monsieur Recchi et vous avez raison, y a traité constant, une coopération renforcée peut-être utilisé ou la coopération structurée permanente dans le domaine de la défense ou s'il faut envisager des coopérations intergouvernementales dans un 1er temps. Tous ces instruments existent et ont été utilisés, vous avez eu raison de le rappeler, Monsieur le Président, Bizet comme pour Schengen ou encore pour le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, nous voulons le faire dans un esprit résolument européen en donnant envie à tous nos partenaires d'avancer. Résumé : notre démarche à une progression vers une Europe fédérale, monsieur ne me paraît pas faire totalement justice à la qualité et à l'originalité du projet que nous portons en parallèle, nous devons aussi préserver le fondement de ce que nous partageons toujours à 28 aujourd'hui, demain, à 27 bien à bien entendu au marché unique, mais aussi à l'État de droit monsieur Ouzoulias dans une Europe refondée, nous devons nous assurer de disposer d'instruments plus efficaces pour assurer son respect au sein de l'Union européenne elle-même, en veillant à ce que la cohésion de notre union soit autant une cohésion démocratique, économique ou budgétaire. Je souhaite revenir sur les conventions démocratiques

car ces conventions joueront un rôle essentiel pour que la refondation de l'Europe que nous appelons de nos voeux puisse voir le jour, soyons clairs, nous ne pourrions atteindre nos objectifs et plusieurs d'entre vous avez relevé qu'ils étaient ambitieux s'il ne suscitait que l'indifférence des Européens et d'abord en ce qui nous concerne, des Français, il serait absurde de vouloir refonder l'Europe sans eux ou en se contentant de leur demander d'un d'exprimer un avis. Par une procédure simpliste de oui ou non, à l'issue d'un long processus de négociation, au contraire, nous voulons donner la parole aux Français et partout aux Européens les écouter et leur donner l'occasion de dire là où l'Europe répond à leurs attentes. Là où elle est déçoit là où elle manque d'ambition et ce qu'il voudrait qu'elle puisse faire pour. Parfois la elle là où elle devrait intervenir moins. Jean-Yves Le Drian, vous a présenté les grandes lignes du dispositif des débats publics, physiquement comme en ligne dans les institutions mais aussi dans les universités, les lieux de culture, les entreprises, les associations et avec tout ce désamour retransmis de l'Europe aux opposants les plus déterminés qui voudront s'exprimer car l'Europe nous concernent tous, elle insiste sur la nécessité de donner la parole à tous nos concitoyens, et pas uniquement aux habitants de Paris et des grandes villes, nous voulons entendre les Français au plus près des territoires en mobilisant les acteurs de terrain. élus de cette assemblée, en particulier, élus locaux, chefs d'entreprise, responsables syndicaux, membres du secteur associatif. Nous voulons faire tout cela au cours du 1er semestre 2018 avec les pays qui le souhaiteront en trouvant le bon équilibre entre le partage de principes et de moyens d'action commun et une dose nécessaire de flexibilité pour chaque État-membre. Vous avez évoqué, messieurs les présidents, Cambon et Bizet l'importance du Brexit. Et je salue le rôle joué par le groupe de suivi mis en place par vos 2 commissions. S'agissant particulièrement des questions de défense, Jean-Yves Le Drian, a souligné à la fois notre détermination à poursuivre. Nos relations étroites avec le Royaume-Uni, notamment dans le cadre auquel nous sommes très attachés, du traité de l'enclave, mais il a rappelé aussi la nécessité de respecter strictement les principes que nous nous sommes donnés à 27 et notamment l'unité du canal de négociation, j'en profite pour saluer comme l'a fait le président Bizet le travail difficile que réalise Michel Barnier. Et la nécessité que les projets cette des progrès satisfaisants soit enregistrée sur les 3 sujets prioritaires définis par le Conseil européen, droits des citoyens frontière règlement financier avant d'élargir le Champ des discussions et d'évoquer nos relations futures ou ce qui est lié une éventuelle période transitoire. Le discours de Madame May à Florence, a présenté des avancées sur ce dernier aspect, mais elles, elles ne se sont pas encore traduites par des progrès dans la négociation des 3 priorités, notamment sur le règlement financier j'ajoute que cela ne veut pas dire qu'à titre national, nous restions inerte ou bien au contraire, car de nombreux secteurs sont sensibles, vous avez évoqué la défense il y en a beaucoup d'autres, la pêche, par exemple, nous nous préparons donc et nous serons prêts le jour où la négociation de l'accord futur s'engagera, je voudrais maintenant répondre brièvement à quelques unes des interventions qui ont concerné des sujets plus sectorielles. Madame et le président Bizet et vous avez cité Erasmus oui Erasmus est l'un des succès européens les plus marquants, parce qu'il a changé la vie quotidienne des jeunes européens, pour l'instant, essentiellement des étudiants, nous voulons en effet aller plus loin et Ralph doit être généralisée pour les étudiants, mais aussi pour les apprentis qui sont encore trop peu nombreux à en bénéficier plus largement, nous voulons qu'en 2024 la moitié d'une classe d'âge européen d'Européens est passé au moins 6 mois dans un autre pays que le sien avant ses 25 ans, cela passe aussi par un processus de la Sorbonne pour que les jeunes puissent passer d'un système d'enseignement secondaire à un autre. Sur l'Erasmus des représentations nationales, vous me permettrez monsieur Gattolin de ne pas me prononcer et de respecter ainsi scrupuleusement la séparation des pouvoirs. Mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier pour le grand honneur que vous m'avez fait en me donnant cette opportunité de m'adresser à vous, cet après-midi, ici devant le drapeau tricolore et devant le drapeau européen, Monsieur Guillaume, le gouvernement sait pouvoir compter sur le Sénat et sur les sénateurs pour donner corps au quotidien et au plus près des territoires à ce débat indispensable sur l'Europe, je veux enfin vous dire toute la fierté que je ressens en tant que ministre et en tant qu'européenne convaincue à ce que la France porte à nouveau le débat sur l'Europe et soit à nouveau au coeur du débat européen, notre place n'est nulle part ailleurs, je vous remercie. 30 projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations 45, les questions d'actualité au gouvernement à 17 heures 45 suite éventuelle du projet de loi, la séance est levée.